La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème : « La contribution des politiques d'appui aux collectivités à l'aménagement et la cohésion des territoires.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

s'il est un débat qui a toute sa place dans notre hémicycle, le Sénat étant le représentant des territoires dans leur diversité, c'est bien celui des politiques d'appui à l'aménagement et la cohésion des territoires.

Dans les faits, nous avons tous pu constater et faire remonter les retards à l'allumage liés à la mise en place de l'Agence nationale de la cohésion des territoires Cette structure reste un bel horizon. L'appui que recherchent nos territoires n'est pas que financier : le soutien par l'intermédiaire des fonctions support, l'ingénierie notamment, est au coeur d'une meilleure conception de l'aménagement local. Vous le savez, les écologistes aiment penser global et agir local. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires a souvent dénoncé les mouvements de recentralisation et de déconcentration qui perturbent l'autonomie de nos territoires.

Plus qu'un pacte de gouvernance, c'est une nouvelle vision de l'organisation territoriale dont nos villes et nos régions ont besoin, une organisation bâtie et pensée avec elles et pour elles, pour accompagner au mieux leurs politiques d'aménagement et de cohésion. Or les politiques d'appui aux collectivités sont encore trop centralisées. L'ambition d'une décision et d'un soutien plus locaux, moins verticaux, semble s'éloigner. Ce débat renvoie à la réalité de tous les jours, à la vie concrète et sensible des Français au quotidien

Madame la présidente,

de concilier intérêt local et intérêt général. La métropolisation poursuivie sous ce quinquennat aura renforcé les distorsions, concentrant les financements et les pouvoirs dans les centres urbains.

le désengagement de l'État de sa responsabilité première d'aménageur. J'en veux pour preuve la volonté de l'exécutif de se dessaisir des routes ou des petites lignes ferroviaires, toutes les infrastructures qui s'articulent en réseau. Le Sénat l'a refusé au nom de l'unité du patrimoine et de la nécessité d'un État qui relie les territoires, plutôt qu'il ne les segmente.

En réalité, cette stabilité n'est même qu'illusoire, puisqu'elle ne prend pas en compte l'inflation. Qui pis est, l'autonomie financière et fiscale des collectivités locales a été largement remise en cause par la nationalisation de la taxe d'habitation,

si utile pour nos territoires qu'il conviendrait de pérenniser. Les politiques de soutien aux collectivités dans le domaine de la construction ont également été revues à la baisse, puisque l'État s'est progressivement désengagé de la production de logements abordables.

que par un appui spécifique aux collectivités, elles passent aussi par une déclinaison efficace de politiques nationales adossées sur le respect des droits de l'ensemble de nos concitoyens, notamment au titre du principe d'égalité devant le service public.

puisqu'elles ne servent qu'à gérer la pénurie et masquer le fait que des pans entiers de notre économie ont été privatisés au détriment de l'intérêt général. Il faut une loi d'aménagement du territoire reposant sur trois piliers

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le débat qui nous réunit aujourd'hui porte sur une thématique chère à la Haute Assemblée : la contribution des politiques d'appui aux collectivités à l'aménagement et la cohésion des territoires. Comment garantir le développement de tous les territoires sans risquer une rupture d'égalité entre ces derniers ? Comment favoriser la cohérence territoriale, tout en prenant en compte les circonstances locales ? Voilà quelques-unes des interrogations que nourrissent nos échanges.

Il reste néanmoins à voir si sa traduction sur le terrain confirmera la démarche initiale. Les politiques d'appui en faveur des collectivités ne sont pas le remède à tous les maux.

Il n'est pas rare qu'une municipalité ne dispose pas des ressources humaines nécessaires ou de services suffisamment étoffés pour répondre aux nombreux appels à projets nationaux. C'est pourquoi je m'interroge sur les solutions concrètes que peut apporter le préfet de département, en qualité de délégué territorial de l'ANCT.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues,

Sans revenir sur le Congrès des maires, il me semble primordial de rappeler que la confiance entre l'État et les collectivités repose, d'abord, sur la clarté et la stabilité de la norme, ensuite, sur la péréquation entre les territoires pour garantir la solidarité nationale, enfin, sur l'accompagnement humain, juridique et financier pour les territoires les plus défavorisés. C'est sur ce dernier point qu'il nous semble important d'insister. S'agissant de l'administration déconcentrée, nous connaîtrons pour la première fois, à la veille des échéances électorales, une progression des effectifs de l'État à l'échelon des départements, après une diminution constante depuis 2007 ... Le groupe du RDSE s'en réjouit vivement.

Cela défie toute logique, alors que son expertise est précieuse au regard de l'ensemble des enjeux d'aménagement du territoire et qu'il existe une véritable carence d'ingénierie au sein d'un grand nombre de collectivités. Cette cure d'austérité doit cesser. madame la ministre, le groupe du RDSE a promu la création, voilà deux ans, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui monte progressivement en puissance. Cela ne va pas assez vite et il faut comprendre l'impatience des élus après des décennies d'abandon de la politique d'aménagement du territoire et de la priorité octroyée aux métropoles, qui ont ainsi pu concentrer les richesses, les emplois et les services. Si l'on progresse enfin vers une logique de guichet unique et le décloisonnement des services administratifs de l'État, un effort particulier sur l'ingénierie territoriale

de 20 millions d'euros ne peut nous satisfaire, sachant qu'elle correspond à un total de 750 projets en 2021 et qu'environ la moitié de cette enveloppe est en réalité dédiée à des prestations réalisées par le privé. par le privé. La création de l'ANCT avait également pour objectif de mettre un terme à la concurrence entre les territoires par le recours aux appels à projets. Nous ne nions pas l'intérêt des programmes menés par l'État, mais ils excluent encore les collectivités n'ayant pas les ressources pour y répondre et monter les dossiers.

Enfin, je tiens à souligner que, sur le terrain, nous constatons des problèmes de cohérence quant à l'identification des territoires bénéficiaires de certains programmes d'État offrant un accompagnement en ingénierie. En Occitanie, par exemple, seules 225 communes ont été labellisées dans le cadre du programme Petites Villes de demain. La région a mis en place des contrats Bourgs-Centres dès 2017, qui concernent toutes les communes ayant des charges de centralité, à savoir les communes dites pôles de services supérieurs et intermédiaires, celles de plus de 1 500 habitants possédant une fonction de pôle de services de proximité et celles de moins de 1 500 habitants, souvent d'anciens chefs-lieux de canton, qui offrent des services essentiels auprès des zones rurales de faible densité démographique. Cela représente en tout 501 communes. Que fait-on des oubliés de l'action territorialisée de l'État ? Nous appelons donc à plus de lisibilité quant à l'identification des bénéficiaires de ces programmes et à une déconcentration et un renforcement des moyens de l'ANCT, notamment sur le terrain, pour soutenir les collectivités qui en ont le plus besoin dans l'exercice de leurs compétences. Madame la ministre, les collectivités territoriales n'attentent de l'État qu'un accompagnement effectif, leur permettant de maintenir des bassins de vie, de faciliter l'accès aux services publics, de concrétiser leur droit à se développer- en somme, l'équité et la cohésion territoriale ! La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mardi dernier, je regrettais en tant que président de la commission des finances que nous nous privions d'une séquence budgétaire de mon point de vue toujours utile. Aujourd'hui, une nouvelle séquence s'ouvre, avec un débat thématique auquel je souhaite contribuer en tant que rapporteur spécial de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». En abordant ce débat, il ne vous surprendra sans doute pas que je revienne avant tout sur la question de l'autonomie financière des collectivités

Par ailleurs, la réforme des impôts de production se traduira par le remplacement de recettes foncières par une dotation, certes évolutive, de l'État pour un montant équivalent à 3,2 milliards d'euros en 2021. Au total, après la réforme de la taxe d'habitation et celle des impôts de production, la part des recettes fiscales sur lesquelles les collectivités locales exercent un pouvoir de taux ou d'assiette s'élèverait à environ 62 % pour les collectivités du bloc communal, 33 % pour les départements et 10,6 % pour les régions. De ce point de vue, on observe que, dans le total des ressources financières des collectivités, les ressources issues de la fiscalité directe locale diminuent année après année- force est de reconnaître que cela ne date pas d'aujourd'hui -, au profit de transferts financiers de l'État.

Revitalisation des centres-bourgs ou autre, il faut parfois jongler avec des critères relativement rigides. Madame la ministre, au mois de mai 2021, la Cour des comptes indiquait que « ces approximations dans les appellations et les concepts [étaient] en fait révélatrices de l'imprécision de la stratégie de l'État ». En voulant En voulant mettre en place une politique d'encadrement budgétaire des collectivités, l'État organise l'aménagement et la cohésion des territoires, en ne laissant à ces dernières qu'une marge de manoeuvre réduite. Dans l'instruction générale Dans l'instruction générale du 2 février 2021 relative à la composition et règles d'emplois des dotations et fonds de soutien à l'investissement en faveur des territoires en 2021, on trouve d'ailleurs des consignes très claires de mobilisation de ces dotations au bénéfice des différentes démarches partenariales impulsées par l'État- agenda rural, Territoires d'industrie, Petites Villes de demain, Action coeur de ville -,

Si l'on peut parfaitement comprendre et admettre que des concours financiers soient fléchés par l'État sur des priorités définies par lui, encore faudrait-il que des fonds suffisants soient libres d'emploi pour permettre aux élus d'engager des politiques publiques d'aménagement adaptées en fonction de leurs territoires, politiques qui font souvent l'objet d'engagements électoraux. Paradoxalement, la gestion des collectivités territoriales est aujourd'hui de plus en plus jugée par nos concitoyens à l'aune de politiques publiques qui sont, en réalité, largement décidées par l'État. Madame la ministre, sur ce sujet, n'est-il pas temps de réguler et de trouver le bon équilibre entre subventions fléchées, qui peuvent se comprendre, et financements libres d'emploi, totalement nécessaires ? La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, on ne saurait bien évidemment minimiser la contribution des politiques d'appui de l'État, qui est primordiale pour les collectivités, surtout et avant tout en période de crise. Pour autant, nous nous devons d'interroger l'existant, pour que cette action soit efficace et pérenne. Ainsi, à l'heure des grandes transitions et compte tenu des évolutions de plus en plus rapides, quelles sont les attentes des collectivités, mais aussi leurs perspectives ? Quelle est, par ailleurs, la stratégie de l'État en matière d'approche contributive

Sur ce sujet, nous ne pouvons bien évidemment pas passer à côté de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en 2020, sous l'impulsion de la proposition de loi

Bien évidemment, ceux-ci savent se prendre en charge, mais ils se heurtent aux complexités et enchevêtrements des dispositifs actuels. À ce titre, je salue la volonté de mettre en place un fonctionnement efficace et partagé, avec, à la fois, un rôle de l'ANCT en matière de coordination des opérateurs nationaux avec lesquels elle a contractualisé des préfets de département. Il faut particulièrement préserver les financements de ses partenaires, sans quoi son efficacité sera réduite. Les élus sont satisfaits de disposer de ce guichet unique, et les comités locaux de cohésion territoriale de l'ANCT doivent maintenant pouvoir pleinement jouer leur rôle pour s'inscrire dans le dispositif et adopter une approche différenciée. L'ANCT doit permettre une démarche transversale : partir de la réalité vécue par les villes et faire en sorte de leur donner les bons outils en mobilisant toutes les parties prenantes pour faire du « cousu main », mais également offrir une capacité de coordination des ressources disponibles dans la durée, favoriser le partage d'expérience et la montée en compétences des bénéficiaires. L'innovation publique locale ne doit pas être découragée par un plan national au périmètre préétabli par l'État. L'ANCT, en fluidifiant et rationalisant l'existant, doit permettre aux territoires moins denses de se développer par des projets propres, sans voir leurs potentialités aspirées par d'autres territoires plus aguerris. En tout état de cause, une contribution efficace des politiques d'appui en matière d'aménagement et de cohésion passe avant tout aujourd'hui par la contractualisation, en ce qu'elle offre de cohérence avec la prise en compte de la décentralisation et des spécificités locales.

et une unification des dispositifs de contractualisation existants entre l'État et les collectivités territoriales. On ne saurait oublier, madame la ministre, les zones de revitalisation rurale, les ZRR, pour lesquelles nous attendons avec impatience la mise en place du groupe de travail. Si les CRTE permettent d'améliorer la lisibilité de l'action publique, la temporalité des programmes est primordiale. Il faut concilier court et long termes, s'adosser aux projets de territoire et pérenniser les projets lancés. ces temporalités doivent être alignées sur la durée d'un mandat, j'insiste particulièrement sur ce point. De même, une approche en péréquation doit pouvoir être envisagée. Enfin, la question de la mutualisation des actions entre les communes et l'intercommunalité est importante. La crise sanitaire et économique que nous subissons encore aujourd'hui a mis en exergue le rôle clé joué par les communes et les EPCI, aux côtés de l'État et des régions, pour gérer l'urgence. Il s'agit à présent de pérenniser cette coopération pour conforter la reprise et renforcer économiquement les territoires dans les années à venir. Quelle est la position du Gouvernement sur ces points ? En conclusion, toute politique d'appui se doit de proposer un cadre souple, capable d'intégrer les évolutions de la décentralisation et la progression des capacités des collectivités locales. C'est par le prisme de cette approche que nous nous permettrons de poser un regard critique sur votre engagement et votre capacité d'action sur le sujet, madame la ministre, et que nous jaugerons une nouvelle politique contractuelle qui se doit de donner de la lisibilité aux collectivités et de garantir l'engagement de l'État dans la durée.

un certain nombre de préfets ont tendance à ne plus traiter qu'avec les présidents d'EPCI, laissant de côté les maires qui n'y sont pratiquement plus associés et qui manquent par conséquent totalement d'information. Tout ou presque se passe comme si ces préfets avaient perdu leur boîte mail Si cette pratique devait perdurer et se généraliser, ce serait alors la fin du couple maire-préfet, si cher au Président de la République. J'ose espérer, madame la ministre, que vous saurez le rappeler à qui de droit sujet a trait au déploiement des conseillers numériques sur le territoire national. À la faveur du plan de relance, l'État a décidé de consacrer 250 millions d'euros en 2021 pour soutenir la lutte contre l'illectronisme. Cette initiative, pilotée par l'ANCT, répond à une attente d'un grand nombre de nos concitoyens et je la salue, comme il se doit. salue, comme il se doit. Les premiers conseillers sont à présent sur le terrain, mais déjà se posent deux questions. La première interrogation porte sur le financement des emplois à l'issue de la période contractuelle prévue. Elle est importante, car elle conditionne grandement la fidélisation des agents recrutés, qui pourraient être tentés de saisir des opportunités plus pérennes. Madame la ministre, pouvez-vous vous engager sur la prise en charge par l'État de la poursuite de ces contrats au-delà de la durée prévue de trois ans ?

lorsque cette formation a lieu dans un endroit éloigné- parfois très éloigné -du lieu de travail et qu'elle occasionne des frais pouvant aller jusqu'à 6 000 euros ? Ce sont des sommes importantes pour les petites communes qui se sont engagées aux côtés de l'État pour favoriser l'inclusion numérique au plus près des territoires.

Ces agents, qui remplissent leur fonction avec compétence et efficacité, se trouvent ainsi privés d'une prolongation de leur contrat, au motif qu'ils ne sont plus prioritaires. C'est d'autant plus dommageable que certains sont parfois proches de l'âge de la retraite et qu'ils ne trouveront aucun autre emploi. Gouvernement envisage-t-il de demander à Pôle emploi d'appliquer la nouvelle réglementation avec souplesse ? Il conviendrait de tenir compte de la situation particulière des agents de plus de 50 ans, voire de plus 60 ans, en fonctions au moment de l'évolution réglementaire.

les dépôts de recettes dans son réseau départemental. Elle demande aux régisseurs de les déposer dans un bureau de poste ou une agence postale. C'est ainsi dans le département de la Moselle. Alors que ces dépôts faisaient l'objet d'un recomptage contradictoire en présence à la fois du régisseur et de l'agent des services fiscaux, la procédure a changé avec La Poste. La recette est désormais recomptée ultérieurement au dépôt. En cas de résultat inférieur à la somme déclarée, la différence est automatiquement imputée au régisseur. Cette pratique est pour le moins choquante ! C'est pourquoi je vous demande, madame la ministre, d'user des relations particulières que l'État entretient avec le groupe La Poste

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les collectivités territoriales ont été particulièrement sollicitées pour la gestion de la crise sanitaire. Elles continueront à l'être, sans doute davantage encore avec les défis de la transition écologique. Elles doivent donc être en mesure d'élaborer une conduite stratégique et anticipative de leur développement, afin que celui-ci soit durable et résilient. Cela suppose qu'elles bénéficient d'une ingénierie. Or la présence des compétences est loin d'être équitable et homogène sur l'ensemble du territoire. Les grandes collectivités, qui ont le plus de moyens, ont pu développer leurs propres ressources ou disposer d'une puissante expertise externalisée. À l'inverse, les plus petites, qui disposent de budgets et d'effectifs bien moins importants, notamment en milieu rural, sont dotées de peu de compétences en interne et manquent de moyens adaptés pour mener à bien leurs projets. Elles doivent donc pouvoir compter sur l'expertise et l'accompagnement de l'État.

ceux-ci, tant financiers qu'humains, demeurent insuffisants. Ainsi, pour les collectivités en demande d'ingénierie, il est fait état de 400 projets accompagnés en 2021 et d'une cible de 500 projets en 2022 et 2023.

Par ailleurs, le soutien de l'ANCT n'intervient que dans le cadre des programmes d'action qu'elle pilote. Qu'en est-il des communes qui n'entrent dans aucun des dispositifs, comme les programmes Action coeur de ville ou Petites Villes de demain ? Ces trous dans la raquette laissent pour compte des collectivités en difficulté. En outre, entre les différents dispositifs, les politiques de labellisation ou encore les contrats de ruralité, l'action de l'État en direction des espaces ruraux est en elle-même d'une grande complexité, ce qui rend le soutien en financement et en ingénierie technique peu lisible pour les collectivités territoriales qui peuvent en bénéficier. Il s'agit en somme d'un système absurde, dans lequel l'accès à l'aide de l'État est si laborieux que celle-ci n'est finalement pas à la portée des collectivités qui en ont le plus besoin. Aussi continuons-nous à appeler le Gouvernement à mettre en place une intervention ciblée, prioritaire et renforcée, au profit des territoires les plus en détresse pour identifier et actionner rapidement les leviers potentiels de développement. Enfin, nous tenons à rappeler que la décentralisation ne doit pas être appréhendée comme un désengagement ou un dessaisissement de l'État. Si le déploiement des politiques territorialisées échappe de plus en plus à l'action strictement nationale, le renforcement des pouvoirs locaux ne doit pas pour autant faire perdre de vue le rôle éminemment stratégique qui doit encore être celui de l'État en matière de cohésion et de développement équitable des territoires. À cet égard, on ne peut que regretter on ne peut que regretter le mandat pour rien du haut-commissariat au plan, cette coquille vide qui aurait pu et aurait dû penser la solidarité et la complémentarité entre nos territoires et leur transformation à l'aune du réchauffement climatique. Le développement, indispensable mais anarchique, des éoliennes, concentrées dans quelques régions,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'aménagement du territoire a de tout temps été un enjeu majeur. un défi crucial guide de plus en plus nos politiques publiques, celui que pose le dérèglement climatique. L'aménagement du territoire en tient compte.

Nous avons besoin d'espaces préservés pour notre biodiversité, faune et flore mélangées, et pour notre agriculture. J'ai été interpellé récemment sur un sujet particulier en Loire-Atlantique : le sort du littoral dans la nébuleuse de l'artificialisation des sols. Pour être plus concret, je prendrai pour exemple le pays de Retz, la Côte d'Amour, la Côte sauvage. De nombreux littoraux français rencontrent les mêmes problématiques.

inondations plus fréquentes et tempêtes aux violences inouïes, comme Xynthia en 2010. Cette commune accueille par ailleurs un flux de population qui s'est accentué dans les dix-huit derniers mois. Depuis le début de la pandémie en effet, les grands centres urbains sont délaissés pour la campagne, les petites villes et les littoraux. Le prix du foncier est donc en nette augmentation et les possibilités de construction sont restreintes. Cette flambée des prix complique la capacité des municipalités à agir.

et entraînent même parfois des contresens. Il est évident que l'artificialisation de nos sols doit, à terme, se réduire drastiquement. Cependant, les territoires littoraux ou ruraux doivent pouvoir accueillir de nouveaux arrivants et leur offrir des perspectives économiques, si nous voulons maintenir leur dynamisme.

qui sont sous tension en termes d'espace disponible, avec un foncier dispendieux, peuvent avoir du mal à remplir l'obligation d'un pourcentage minimal de logements sociaux. Quand ils trouvent des solutions raisonnables et équilibrées entre toutes les préoccupations auxquelles ils doivent faire face, les élus locaux sont parfois victimes d'insultes et de menaces, les populations refusant que le charme attractif d'une ville balnéaire soit rompu par l'émergence d'immeubles. Tous les témoignages que j'ai recueillis expriment la même volonté d'une véritable différenciation dans les territoires, pour répondre à leurs besoins spécifiques que les acteurs locaux sont le mieux à même d'identifier précisément. de l'artificialisation illustre parfaitement la nécessité de nous doter de politiques publiques adaptées en fonction des territoires, elle n'est pas la seule. Bien des domaines le prouvent. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la France est riche de ses diversités. Les politiques publiques qui les accompagnent doivent l'être tout autant.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez inscrit à l'ordre du jour de vos travaux ce

Vous m'interrogez sur la manière dont les politiques de soutien de l'État aux collectivités territoriales contribuent à l'aménagement et à la cohésion des territoires. est vrai que l'État considère qu'il a une mission d'appui aux collectivités territoriales : à elles l'aménagement de leur territoire, à lui l'aménagement du territoire national, dans une logique de subsidiarité.

C'est une politique très importante, partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Il ne s'agit pas d'imposer, mais il arrive un moment où c'est

nationale, je précise qu'un certain nombre de départements, comme la Nièvre, les Ardennes ou la Creuse, ont bénéficié d'une augmentation (DGF), et ce malgré la baisse de population de ces trois départements. Par ailleurs, l'État y a lancé des pactes d'aménagement spécifiques.

Un tiers du budget de l'ANCT, soit 20 millions d'euros, est destiné au financement du marché d'ingénierie de l'ANCT, qui permet d'aider les collectivités à concrétiser leurs projets en bénéficiant d'expertises externes

Je précise même que les aides sont gratuites pour les communes de moins de 3 500 habitants et pour les intercommunalités de moins de 15 000 habitants. Les territoires ruraux sont donc particulièrement ciblés, car nous savons bien

Benarroche, nous travaillons aussi sur la métropole Aix-Marseille-Provence. J'espère que nous aboutirons à un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur le sujet.

Nous estimons qu'elles doivent être amplifiées dans les territoires ruraux- cela représente 80 % du territoire et un tiers de la population -, afin de réduire les inégalités territoriales et d'y maintenir la vie. En complément de ce qui existe, un appui

pour tous. Il faut également donner la possibilité aux agriculteurs de diversifier leur production en maintenant les possibilités d'irrigation, et ce avec des préfets développeurs. s'agisse de Petites Villes de demain, de ceux que vous avez mis en place ou de ceux qui permettent la réhabilitation et la rénovation de nos centres-bourgs, sont nécessaires pour l'urbanisation. L'artificialisation des terres doit être différenciée par rapport aux villes et permettre au monde de faciliter la réalisation de maisons individuelles. L'accès à France Services doit être généralisé dans tout le pays. Le Gouvernement est-il favorable à la mise en place de ZRR mieux ciblées dans les territoires ruraux après 2022 ?

Cet appui va bien au-delà du seul soutien financier : c'est la mise à disposition de tous les moyens, humains, techniques ou juridiques, nécessaires à l'aménagement du territoire. La semaine dernière, j'ai souligné en commission de la culture le défaut d'ingénierie dont pâtissent nos communes.

Ainsi, les petites communes n'ont guère d'administration ni même de cabinet pour appuyer leurs élus. Elles ne peuvent pas bénéficier d'administrateurs territoriaux. Le seuil démographique constitue un frein à des recrutements nécessaires, comme l'a souligné un rapport d'information publié l'année dernière. dernière. Il estimait que 30 000 communes ou intercommunalités ne disposaient pas des moyens suffisants pour organiser leurs propres services d'ingénierie. Par ailleurs, les plus petites communes doivent être associées aux politiques mises en place, comme on le voit dans le développement des contrats associant l'État aux intercommunalités. telles associations sont nécessaires, les communes ne doivent pas être noyées. Nous veillerons à ce que tous les maires soient impliqués, afin que ces contrats profitent à tous.

J'en viens aux mécanismes de péréquation, qui loin d'être optionnels pour un territoire comme le mien, sont au contraire vitaux, en particulier pour les conseils départementaux, qui sont sous perfusion totale et qui connaissent un reste à charge insupportable. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour que les communes les moins peuplées, les plus immergées dans la ruralité, celles qui ont le moins de ressources, bénéficient concrètement de ces politiques et disposent des moyens suffisants pour réaliser leurs projets ? La parole est à Mme la ministre. Madame la

M. Guillaume Gontard. Madame la ministre, depuis vingt ans, les gouvernements successifs ne cessent de rogner sur l'autonomie fiscale des collectivités locales. En la matière, le Gouvernement a battu tous les records avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. de cette réforme, ce sont plus de 30 % de leurs recettes que les élus locaux ne peuvent dorénavant plus moduler ! Alors que s'opérait cette recentralisation fiscale, les transferts de compétences de l'État vers les collectivités se poursuivaient, creusant un fossé toujours plus béant entre les moyens des collectivités et leurs responsabilités. Tout à sa stratégie d'endiguement de la dépense publique, l'État continue de couper le robinet en direction des collectivités, tout en insistant sur leur rôle essentiel dans tous les domaines : relance économique, gestion de la pandémie, transition écologique, Reconnaissons tout de même que le Gouvernement innove en matière de contrôle fiscal, en allant jusqu'à contraindre les collectivités dans leur capacité à moduler les taux des impôts locaux. Cette disposition n'a pas fait grand bruit lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. de la fin de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes ne pourront plus faire évoluer le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires comme elles le souhaitent. En effet, de manière assez peu compréhensible, ce dernier sera lié désormais au taux de la taxe sur le foncier bâti. Pour de nombreuses communes pourtant, en particulier pour les communes touristiques, cette ressource est essentielle. Elle a le double mérite de cibler les ménages les plus aisés propriétaires de résidences secondaires et de lutter contre la sous-occupation des logements.

est établi entre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière, on voit bien qu'il vise à protéger les intérêts des multipropriétaires. Je trouve cela particulièrement dommage. La

Ce problème va, puisque cette proportion n'était que de 7 % en 2012. Les raisons en sont multiples- de l'incapacité des gouvernements successifs à anticiper la démographie médicale sur le moyen et le long terme à la vague massive de départs à la retraite de médecins généralistes, en passant par l'absence de mesures radicales, de peur de froisser un lobby médical politiquement sensible. Certes, des mesures ont été prises et des solutions mises en place, mais elles relevaient plus de l'homéopathie que de la médecine d'urgence. Même l'égalité d'accès aux soins, dont la France pouvait, par le passé, s'enorgueillir, se délite : on compte un médecin pour 400 habitants dans les Alpes-Maritimes et moins d'un médecin pour 1 000 habitants dans l'Eure ou en Seine-et-Marne. Les gens sont-ils plus malades à Nice, Cannes ou Antibes qu'à Évreux ou Melun ? notre devise républicaine, issue de l'article 2 de la Constitution, est bousculée. Si l'on ajoute à ce constat statique qu'un tiers des médecins généralistes ont plus de 60 ans, on ne peut qu'appréhender l'avenir.

le temps des rapports, des constats, des concertations et des mesurettes doit laisser place à un plan Marshall. Ayez de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, pour sauver la carte sanitaire française et, enfin, entendre les oubliés de la santé ! La parole est à Mme la ministre.

Pour y faire face, les communes, les EPCI, les départements ou les régions ont augmenté considérablement leurs dépenses de fonctionnement, en embauchant du personnel médical, en achetant en plus grande quantité des produits d'hygiène et d'entretien, en investissant dans du matériel de détection- le fameux capteur de CO2 -, de protection- les masques -ou encore de prévention- les purificateurs d'air.

Ce même rapport met également en exergue les inégalités d'investissement selon les collectivités, avec un recul net du montant investi pour le bloc communal. Dans un département comme le mien, qui compte 890 communes, vous comprendrez, madame la ministre, que je sois régulièrement interpellé par les élus. Ces derniers s'inquiètent des hausses annoncées pour 2022 des matériaux et matériels pour le BTP, alors même que ces matériaux ont déjà subi une augmentation de 15 % à 20 % en 2021.

en priorité appel à l'État et 18 % au secteur privé. Surtout, moins de 50 % des répondants connaissent l'ANCT. Parmi eux, 22 % seulement ont fait appel à ses services.

des budgets départementaux. La parole est à M. Bruno Rojouan. Avec la crise sanitaire, certains de nos concitoyens ont fait le choix de se confiner hors des grands centres urbains et ont ainsi redécouvert les charmes et la qualité de vie des zones rurales et des villes moyennes. Dans certains départements comme l'Allier, nous assistons depuis quelques mois à des ventes de biens qui ne trouvaient pas preneurs. Les nouveaux arrivants sont souvent de jeunes couples d'actifs cherchant à s'éloigner des métropoles et à acquérir une résidence au vert. Ces nouvelles populations sont une chance pour redynamiser la démographie déclinante des territoires ruraux, à condition bien sûr de leur permettre d'y rester par une politique d'attractivité renforcée. Madame la ministre, les territoires dont nous parlons ont de véritables besoins. Ces besoins concernent tout d'abord les infrastructures de communication, puisque de multiples chantiers de réseaux ferrés et routiers doivent encore être menés et la couverture en réseau 4G améliorée. Dans ce domaine, la signature du New Deal mobile a contribué à des avancées, mais ce plan n'a pas su répondre à tous les enjeux du développement numérique mobile et des zones blanches persistent.

concernent la revitalisation des centres-bourgs, enjeu majeur d'une reconquête vivante. Un an après le lancement du programme Petites Villes de demain, un bilan d'étape doit être mené. Madame la ministre, vous le savez, les territoires ruraux se battent chaque jour pour attirer de nouvelles populations. Le soutien de l'État doit être plus puissant. Force est de constater que beaucoup reste à faire en la matière. La parole est à Mme la ministre.

le rôle de nos collectivités dans la gestion des déchets est central. Pour atteindre des objectifs environnementaux ambitieux, il est aujourd'hui nécessaire d'agir pour réduire les déchets à la source, donc d'assister les collectivités dans la mise en place de dispositifs innovants. Le Grenelle de l'environnement prévoyait la possibilité d'inclure une part variable incitative dans les taxes ou redevances d'enlèvement. Cet objectif est loin d'être atteint aujourd'hui, compte tenu des contraintes de mise en oeuvre du dispositif dans les zones urbaines denses, où la part importante de logements collectifs rend la mesure individuelle du tonnage des déchets opérationnellement complexe. Plusieurs collectivités ont imaginé un dispositif de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) incitative à une échelle collective. Ce scénario repose sur l'instauration d'une TEOM incitative basée sur plusieurs flux de déchets ménagers et assimilés, mesurés collectivement par secteurs. Ces secteurs, qui peuvent être des communes, des quartiers ou des îlots, seraient définis par délibération, la collectivité territoriale évaluant notamment l'échelle la plus pertinente. La philosophie de ce scénario novateur repose sur des dynamiques collectives. Elle constitue un élément moteur des changements de comportement,

La loi prévoit que la redevance incitative peut être calculée au niveau d'un bâtiment- immeuble ou maison individuelle -, dans la mesure où il est possible de calculer la quantité de déchets produits à cette échelle. Élargir le calcul de la redevance à tout un quartier pourrait dénaturer l'objet même du calcul. En effet, la collectivité calculerait une redevance pour tout le quartier et la répartirait à parts égales entre les foyers. Cette méthode évidemment les ménages les plus économes et avantagerait ceux qui rejettent davantage de déchets. Par ailleurs, cette proposition poserait des difficultés d'application : le maillage serait complexe à appréhender pour les services fiscaux et les dégrèvements

Alors que, dans certains territoires, les règlements départementaux ont été élaborés avec pragmatisme et bon sens, dans d'autres, comme dans le département de la Seine-Maritime, ils sont devenus une énorme épine dans le pied des élus. Pour certaines communes, le manque de foncier pour installer des bâches ou des réserves d'eau enterrées rend son application impossible. Pour d'autres, le débit d'eau est insuffisant pour installer des poteaux incendie. Pour toutes, ce sont des dépenses démesurées, absorbant parfois jusqu'à la totalité du budget d'investissement du mandat, pour s'y conformer. Sans parler des bureaux d'études non agréés par l'État qui jouent de cette situation pour faire monter les enchères. des permis de construire ne peuvent être délivrés et des aménagements sont empêchés, renforçant le sentiment d'abandon d'élus de milieux ruraux et l'idée que l'on veut asphyxier les petites communes pour les faire disparaître.

Quels accompagnements financiers pouvez-vous envisager pour soutenir les communes ? En Seine-Maritime par exemple, la part de la DETR consacrée à la défense incendie est passée de 1 %

et plusieurs autres sénateurs demandant que le Gouvernement remette un rapport au Parlement au plus tard le 1 juillet 2022, afin d'évaluer la mise en oeuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l'incendie,

Mme Évelyne Perrot. Madame la ministre, ma question porte sur la relation entre l'aérien et les territoires. Derrière la lutte entre l'« aviation » et l'idée en vogue du voyage de revanche après la pandémie, n'oublions jamais un fait essentiel la France dispose d'un pouvoir de marché sur la moitié de la flotte aérienne mondiale, ce qui lui permet d'agir positivement pour la planète et pour les territoires. Des milliers d'emplois et d'entreprises sous-traitantes s'impliquent dans la transition verte de ce secteur haut de gamme. C'est un stimulant pour des formations très qualifiées et l'élévation du niveau du niveau scientifique, dont notre pays a tant besoin. Économiquement, c'est tout un écosystème- aéroports, compagnies aériennes, contrôleurs aériens -qui doit travailler dans le même sens. soulevés. Premièrement, nous fabriquons des avions de plus en plus sobres sans bénéficier de filière pour y incorporer des biokérosènes, dits de deuxième génération, sans ponction sur l'agriculture destinée à l'alimentation. nous risquons de prendre du retard par rapport à nos voisins allemands sur les e-kérosène fabriqués en capturant du CO2. Deuxièmement, 90 aéroports devront investir lourdement pour verdir leurs opérations au sol et préparer l'approvisionnement des avions en nouveaux carburants ou en hydrogène. Il faut combler leurs pertes de recettes dues à la pandémie plutôt que de les inciter à augmenter des prélèvements sur des compagnies aériennes en grande difficulté. je m'interroge sur le développement des petits avions électriques. Avant tout, renouvelons la flotte d'environ 6 500 petits avions bruyants et polluants qui servent à la formation des écoles de pilotage. Un soutien limité de l'État permettrait un gain considérable en décibels pour les riverains. Les pertes de taxes sur les nuisances aériennes bloquent les financements de travaux d'insonorisation, alors que le fret aérien se développe avec des vols de nuit. Or nos concitoyens sont de plus en plus sensibles au bruit. Sur ces trois points, qu'envisage le Gouvernement ? La parole est à Mme la ministre. Madame la sénatrice, le Gouvernement a mené une politique particulièrement proactive de soutien au secteur aérien. Ainsi, dans le cadre du plan de relance, 1,57

il faut savoir que les petits avions électriques ne sont aujourd'hui pas produits en France. Nous centrons donc notre soutien sur la recherche et développement, la R&D, pour faire émerger une filière française de petits avions électriques et hybrides. viens aux conséquences de la crise sanitaire sur l'équilibre économique des aéroports au cours de la période 2020-2022. Le manque à gagner de taxes sur les nuisances sonores aériennes peut être estimé à 80 millions d'euros. Dans un contexte de difficultés financières extrêmement fortes pour les compagnies, il n'est pas prévu de relever les barèmes de cette taxe. Je suis d'accord avec vous, madame la sénatrice, il est essentiel de permettre la continuité d'une politique publique dont l'objectif est de réduire l'impact des nuisances sonores entraînées par l'activité aérienne sur les populations riveraines. Il se trouve ainsi nécessaire de prendre à brève échéance des mesures visant à faciliter le financement du dispositif d'aide à l'insonorisation aux abords des principaux aérodromes.

Madame la ministre, je le répète, les élus locaux sont très inquiets de la reprise épidémique. Au-delà des enjeux économiques, cette pandémie a révélé les failles de notre société et renforcé encore les fragilités liées aux situations d'isolement social et de précarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nos communes sont à la base de la cohésion sociale et territoriale et elles ont su faire face. L'État se doit toutefois de les accompagnera afin qu'elles disposent de tous les outils leur permettant de renforcer leur action en la matière.

Sur l'hébergement d'urgence, d'abord, un effort certain a été consenti en 2021 et reconduit pour 2022, mais seulement à échéance du mois de mars, date à laquelle des solutions de remplacement doivent être mises en place. Les acteurs locaux demeurent inquiets quant à l'effectivité de ces solutions et craignent une rupture dans l'accompagnement, réduisant la portée du travail d'insertion réalisé. Ensuite, les crédits dédiés au logement social sont prolongés, mais la subvention par logement ne progresse pas, alors qu'une augmentation permettrait de développer la production de logements très sociaux. En outre, la rénovation thermique des logements continue d'être encouragée, mais le reste à charge demeure dissuasif pour certains ménages très précaires. au logement (APL) a été très défavorable aux jeunes ménages et son forfait « charges » n'a pas été rehaussé, alors que les coûts de l'énergie ont flambé. Enfin, les crédits de la rénovation urbaine, bien que promis, peinent à être engagés.

de janvier 2021, à la suite du comité interministériel des villes. Les travaux ont démarré à date dans 328 quartiers du NPNRU, contre 210 l'année dernière. Les effets concrets devraient se voir rapidement sur les territoires.

APL visait bien à réévaluer en temps réel les droits de chacun en fonction de ses revenus. La réforme est neutre normalement pour la majorité des bénéficiaires et conduit même à une augmentation pour près de 18 % d'entre eux, selon les chiffres du ministère du logement. Enfin, en matière de logement social, le Gouvernement se fixe

Pour lever ces questionnements, il est nécessaire de mettre en place une évaluation qualitative de cette politique publique pour objectiver ses impacts, donc ses contributions notamment en matière d'aménagement du territoire et de transition écologique. avez-vous prévu une méthodologie partagée d'évaluation de la mise en oeuvre de ces contrats ? Avez-vous également pensé à des objectifs à atteindre en fonction des attendus du contrat ? Les réunions des commissions DETR dans les départements révèlent souvent les ambiguïtés du financement des CRTE. Ne disposant pas de ligne spécifique, le fléchage prioritaire de la DETR et de la DSIL vers les CRTE inquiète fortement les communes qui ne sont pas dans cette contractualisation, le pouvoir discrétionnaire de l'État sur une grande partie des dotations renforçant cette inquiétude. Les crédits disponibles ne couvriront pas l'ensemble des demandes et les CRTE deviendront une obligation pour les collectivités pour être éligibles Prévus pour une durée de six ans, ces contrats restent subordonnés chaque année aux disponibilités inscrites dans la loi de finances et sont cadencés par la mise en oeuvre du calendrier des travaux et du dépôt des dossiers. Mesurez-vous cette incertitude en matière de prévisions financières ? Même sans incertitude financière, le financement des CRTE risque de gager les crédits DETR et DSIL sur plusieurs exercices. Partagez-vous cette analyse ? La parole est à Mme la ministre.

-, qui a pour but de rendre plus lisibles les rapports entre l'État et les collectivités territoriales, ainsi que de répondre aux projets de territoire en finançant aussi bien

ne freine pas le déploiement des financements de l'État. On compte à date 360 CRTE et 530 protocoles de préfiguration signés. Jusqu'à preuve du contraire,

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème : « Quelle action de la France pour prendre en compte l'enjeu environnemental ? »

Ce volontarisme apparent- , conseil de défense écologique, Convention citoyenne pour le climat -se heurte, dans les faits, aux conclusions sévères rendues, en France, sur l'action trop timorée de l'exécutif en matière environnementale. Je n'en prendrai que deux exemples. dans un jugement récent sur ce qui a été nommé « l'affaire du siècle », le tribunal administratif de Paris a reconnu la responsabilité de l'État français dans la crise climatique et jugé illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'État a également été reconnu responsable de « préjudice écologique

et résilience ». Les paroles ne résistent pas aux faits ! Pour autant, l'État a tous les outils entre les mains. En effet, la réglementation est là pour contraindre,

peuvent encourager les citoyens et les entreprises à adopter des comportements vertueux : je pense aux taxes pigouviennes, au marché des droits à polluer ou encore aux subventions à l'innovation.

des conditions de vie, publiée cette année, moins d'un quart des Français sont prêts à payer plus de taxes sur les carburants, le gaz ou le fioul afin de lutter contre le réchauffement climatique. Les Français attendent surtout de la transparence et de la lisibilité dans l'utilisation des recettes fiscales.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le débat qui nous est proposé cet après-midi est particulièrement vaste. Quelle politique environnementale pour la France ? La question est bonne, mais parle-t-on ici de notre stratégie internationale ou de nos politiques publiques dans La réponse n'est pas tout à fait dans la question ... Néanmoins- nous pouvons au moins insister sur ce point en introduction -, les deux échelles sont totalement liées. Ainsi, notre capacité à tenir, chez nous, nos grands objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou à classer 30 % de nos territoires en réserve de biodiversité, autre engagement engagement international que vous défendez, madame la secrétaire d'État, est une condition absolument nécessaire à la conclusion d'accords internationaux ambitieux. Pour le dire encore plus simplement, après l'échec de la COP26 de Glasgow dans son objectif de crédibiliser un scénario de stabilisation du climat autour d'une

est donc bien loin de l'objectif européen présenté à Glasgow. Cela dit notre difficulté collective à agir à la hauteur de ces enjeux, les intérêts immédiats ou de court terme prenant régulièrement le pas sur l'intérêt général de long terme,

Nous sommes très inquiets de voir encore et toujours les effectifs de ces acteurs se réduire d'année en année. Je le redis, nous devons impérativement engager des moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux, notamment en matière d'animation. que la transition écologique nécessite que des acteurs très divers se parlent et élaborent des stratégies communes, ce qui impose d'organiser leur rencontre et leurs discussions. C'est notamment le cas à l'échelle des collectivités territoriales, où se joue une grande partie de cette transition.

moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en oeuvre ; ils risquent de rester en grande partie à l'état d'intention, alors que c'est à l'échelle de ces territoires, par les décisions prises par les élus locaux, que l'action est essentielle pour préserver la biodiversité et réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, tant celles-ci sont liées à notre vie quotidienne. Ce sont bien nos manières de nous loger, de nous déplacer et de nous nourrir qui ont un impact environnemental. Je suis absolument convaincu que nos concitoyens sont prêts à modifier leurs comportements, mais seulement s'ils ont le sentiment que leur effort s'inscrit dans un cadre cohérent,

La France peut-elle jouer un rôle pour relever le défi qui est devant nous ? Sans hésitation, je réponds : oui ! La France peut jouer un rôle original et déterminant pour hisser les sociétés humaines et l'Europe elle-même au niveau des choix politiques qu'il faut opérer pour se mettre à la hauteur des enjeux. Pour réussir ce mouvement, la France devrait avoir trois ambitions politiques majeures : d'abord, faire de l'écologie une grande question populaire,

pour que l'écologie devienne une grande question populaire, il ne faudrait manquer aucune occasion pour orienter nos politiques vers des mesures plus justes socialement et plus avantageuses, d'un point de vue pécuniaire, pour les catégories populaires. Ainsi, si les décisions politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre étaient accompagnées d'avantages financiers ou fiscaux pour les personnes faisant le choix de changer leurs pratiques en matière de mobilités, l'écologie serait vécue par nos concitoyens

Réseau, ce n'est pas à la hauteur. Enfin, il convient de saisir toute la portée de la décision de la Commission européenne de suspendre le pacte de stabilité et de croissance jusqu'à la fin de l'année 2022.

On pourrait, par exemple, exclure du calcul du déficit public les dépenses d'investissement dans la transition écologique,

quelques nuances, y compris au sein du Gouvernement, dont il convient de prendre acte, mais nous pourrions prendre en considération cette situation assez hétérogène à l'échelle européenne et dégager des marges de manoeuvre pour la conduite de politiques d'investissement audacieuses.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, les dernières années ont assurément été synonymes de prise de conscience de l'enjeu environnemental et, tout particulièrement, de l'urgence climatique, mais les années à venir doivent être celles de l'action.

Traduction législative des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, la loi Climat et résilience visait un objectif de réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, tandis que l'ambition européenne était, dans le même temps, rehaussée à 55 %. avions d'emblée émis des réserves quant à la portée effective de ce texte sur la réduction de nos émissions. Sans même tenir compte de l'objectif révisé, le projet de loi présenté au Parlement ne permettait de parcourir qu'entre la moitié et les deux tiers du chemin restant à parcourir entre les émissions constatées en 2019 et la cible pour

qu'il nous était proposé d'examiner, on trouvait un nouveau budget vert visant à améliorer la lisibilité environnementale du budget de l'État. Si nous ne pouvons que nous satisfaire de sa pérennisation, nous appelons également à une accentuation de sa portée et à une amélioration de la méthodologie de son élaboration 92 % des dépenses sont considérées comme neutres, faute de critères pour en mesurer la portée environnementale. Dès lors, comment atteindre cette ambition rehaussée et compléter les mesures déjà adoptées ? convient de soutenir la logique additive consistant à renforcer la capacité de production d'électricité bas-carbone, en associant énergies renouvelables et énergie nucléaire. (RTE) le souligne pertinemment dans son récent rapport, cette logique est celle qui présente le meilleur bilan climatique de court et de moyen terme. C'est donc celle qui est la mieux à même de nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques pour 2030.

Troisièmement, la question de la tarification du carbone doit être abordée en gardant à l'esprit l'impératif de justice sociale, la nécessaire augmentation du prix du CO2 ne pouvant se faire au détriment des plus vulnérables. L'exemple de l'Allemagne, qui propose une redistribution des recettes de la taxe la baisse du prix de l'électricité ou la mise en place d'un forfait énergie, est éclairant. À l'échelon européen, l'heure est évidemment à l'élaboration d'un robuste mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui protégera notre industrie de l'inévitable augmentation du prix européen du carbone. Nous comptons sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour avancer sur ce dossier et convaincre ceux de nos voisins qui pourraient être les plus récalcitrants.

Elle y dénonce un creusement de l'écart entre nos objectifs climatiques et nos résultats, alors que notre pays devra, en application du, réduire de 47,5 % ses émissions d'ici à 2030 pour respecter ses engagements européens. Elle considère que la France, condamnée pour ses progrès insuffisants en matière de lutte contre la pollution de l'air et de protection de la biodiversité, doit mettre en oeuvre une stratégie globale afin d'accélérer la transition de manière équitable et efficace.

La réduction de l'écart entre nos actions et nos objectifs est d'une importance capitale, au-delà des frontières françaises et européennes. Il y va de la survie du cadre international des négociations climatiques, en particulier de l'accord de Paris.

Toutefois, le succès de cette trajectoire dépendra du respect par les États de leur propre feuille de route. Si la France, l'un des principaux contributeurs de l'accord de Paris, et l'Union européenne ne tiennent pas leurs engagements, quel État le fera ?

a donc un rôle historique à jouer pour protéger l'accord de Paris, seul rempart contre la catastrophe climatique qui s'annonce. C'est un honneur pour notre pays, indissociable toutefois de la responsabilité qui nous incombe. Mes chers collègues, nous devons donc agir en responsabilité et accélérer la transition. J'en suis certain, cette grande mutation, source

elles ne figurent pas, pour l'heure, au centre des débats de l'élection présidentielle. C'est à se demander si tous les candidats ont pris la mesure de la situation ! Permettez-moi donc de rappeler certains faits. L'accord de Paris a fixé en 2015 l'objectif de contenir à 1,5 degré Celsius la hausse mondiale des températures d'ici à 2100 par rapport à l'ère préindustrielle. Or, d'après les évaluations des Nations unies, la somme des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre des États nous conduit vers une trajectoire de 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle

Le respect des engagements pris en 2015, confortés récemment lors de la COP26, nécessite un bouleversement de nos modes de production et de consommation, que l'on peine à entrevoir pour l'instant. Même la crise du covid, qui a mis à l'arrêt la plupart des pays du monde pendant des mois, n'a permis une réduction que de 5,4 % des émissions de gaz à effet de serre. La seule solution est donc d'agir immédiatement et drastiquement. À l'échelle de la France, cela signifie mettre l'économie en ordre de marche. On ne peut se satisfaire du adopté par la plupart des grandes entreprises. On ne peut se contenter de la plantation d'arbres en guise de compensation carbone. Nous devons mettre au coeur de nos politiques et de notre économie la sobriété et l'innovation et prévoir à cet effet des investissements massifs. On sait que les grandes innovations, notamment leur diffusion à grande échelle, ne sont pas attendues avant 2050. Il sera alors trop tard pour inverser la tendance.

Si les dépenses en faveur de l'environnement sont en hausse, 10,8 milliards d'euros du projet de loi de finances initial ont des effets défavorables sur l'environnement et 92 % des dépenses générales demeurent neutres. Or, pour que nos engagements soient tenus, il faudrait que l'immense majorité de nos dépenses soient écologiquement vertueuses. Il faudrait que le secteur public, dans toutes ses composantes, se mette en ordre de bataille. Or la mission « Écologie, développement et mobilité durables » prévoit plus de 5 000 équivalents temps plein en moins sur la durée du quinquennat chez les opérateurs rattachés.

la France accusait un retard de 4 points par rapport à l'objectif européen de produire 23 % d'énergie à partir de sources renouvelables. J'en viens là à un point essentiel à mon sens : fixer des objectifs à long terme, sans échéance à court terme et, surtout, sans sanction n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Le GIEC a réaffirmé, dans son dernier rapport, le caractère indispensable d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre. Je parlais plus tôt de sobriété environnementale. Cette notion doit être prise en compte dans toutes nos prises de décision. Elle doit aussi être promue comme une valeur fondamentale à l'échelle internationale. Les conclusions de la COP26 à Glasgow, de même que l'accord entre la Chine et les États-Unis annoncé lors de cette conférence, ravivent l'espoir d'une action diplomatique à la mesure du défi climatique. Les États-Unis sont responsables de 25 % des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère industrielle. La Chine est responsable de 26 % des émissions mondiales de CO2 actuellement. Ce pays demeure très dépendant du charbon.

Ces chiffres sont d'autant plus inquiétants que les changements de modes de consommation et l'expansion des classes moyennes et aisées ont pour conséquence une croissance exponentielle de l'empreinte carbone et des émissions des ménages. Dans ce contexte, la France doit jouer le rôle de porte-étendard de la cause climatique. Il est normal de demander des efforts aux Français. L'enjeu est global et chacun doit y prendre sa part.

j'évoquerai l'exemple de l'albatros. Magnifique oiseau volant sur les océans, déployant une énergie herculéenne pour nourrir son oisillon- un seul chaque année -, il parcourt des centaines de kilomètres de l'atoll de Midway, où il niche, jusqu'aux régions subarctiques très poissonneuses, où il pêche sa nourriture.

non seulement le coût de la tonte est plus élevé que le produit de la vente de la laine, mais cette dernière n'est pas utilisée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une fibre textile. Elle est pourtant naturelle, chaude, douce, isolante, légère, bactéricide, biodégradable, donc noble. À la vérité, est-il encore tenable de faire venir par container, en provenance d'Asie ou d'ailleurs, des vêtements qui rejetteront en permanence des microfibres plastiques dans l'environnement ? Celles-ci sont déjà présentes partout sur terre, aussi bien dans les eaux de l'Arctique que dans les glaces de l'Everest ou dans l'air au Pic du Midi. Elles sont délétères pour nos écosystèmes et pour notre santé. Nous devons produire et consommer localement, ce qui implique une réindustrialisation de notre pays et un changement de nos habitudes de consommation. En favorisant le réemploi, la réparabilité des objets, nous préserverons les ressources. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion sur nos modes de vie et de consommation, sur notre rapport au vivant et au monde. Tant qu'un yaourt parcourra 5 000 kilomètres avant de parvenir dans notre assiette, nous étoufferons sous des canicules. Tant que nous utiliserons sans retenue les glyphosates et autres néonicotinoïdes, les abeilles et les vers de terre disparaîtront, menaçant notre survie même. Tant que la logique de « ma voiture est plus grosse que la tienne » prévaudra, le niveau des océans s'élèvera, les îles Maldives lutteront contre la submersion et seront menacées de disparition.

notamment réparer rapidement les dégâts provoqués par les catastrophes naturelles, à l'instar de celle qui est survenue dans la vallée de la Roya l'année dernière. Dans cette vallée dévastée par une crue inédite, les citoyens se sont heurtés à des freins administratifs et réglementaires inadaptés face à une situation d'urgence. situation devrait être prise dans sa globalité et être encadrée par une loi permettant une reconstruction résiliente et rapide afin de ne pas ajouter des difficultés au traumatisme. Les mesures que nous devons prendre ne peuvent plus être anecdotiques. Elles doivent être à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face. Bien sûr, la contrainte n'est pas la seule méthode à retenir, mais, face au désastre en cours, elle doit avoir toute sa place et être pleinement assumée par les pouvoirs publics. Les citoyens informés sont aujourd'hui prêts à adhérer à des mesures courageuses. Il est temps de leur tenir un discours de vérité. Ceux qui subiront les grands dommages liés à notre inaction sont déjà nés. Nous leur devons de rebâtir un horizon commun de civilisation.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, en 1970, à Chicago, Georges Pompidou, alors Président de la République, définissait la nature « comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'homme de janvier de l'année suivante, il annonçait la création d'un ministère dédié à la protection de la nature. Cinquante ans plus tard, malgré les alertes répétées et un ministère beaucoup plus puissant, notre pays doit poursuivre son action face à l'urgence climatique. Georges Pompidou exhortait la société à « dénombrer les difficultés et à chercher les solutions ». Le constat sur l'enjeu environnemental est largement partagé par les scientifiques et les citoyens. La mondialisation et l'évolution de nos sociétés ont contribué à une dégradation sévère de notre environnement. Il est urgent d'agir. Certaines zones de notre planète sont déjà tellement touchées que les habitants n'ont d'autre choix que de les quitter. Les vagues migratoires qui en résultent, qui sont une réalité, jouent sur les équilibres mondiaux et risquent de s'amplifier dangereusement en raison des enjeux climatiques et alimentaires. En France, des épisodes violents assèchent, détruisent, noient et font souffrir nos territoires. Finalement, notre difficulté majeure est de réussir notre transition en mettant en oeuvre des solutions pragmatiques. Le groupe Les Indépendants-République et Territoires croit en une écologie libérale. Les découvertes scientifiques et techniques diminuant notre impact sur l'environnement sont une grande source d'espoir. Nous devons les soutenir et faire en sorte qu'elles puissent émerger. Notre décarbonation passera par des innovations dans l'industrie, le transport, l'énergie, la construction ou le numérique. Notre consommation doit être placée sous le signe de la sobriété énergétique et de la circularité.

Je n'évoquerai qu'un seul exemple : la stratégie. Notre souveraineté alimentaire est en jeu. N'opposons pas l'écologie au reste du prisme : la réussite réside dans une prise en compte globale. À l'échelon national, deux axes se dessinent. part, ce que l'État fait et décide. À cet égard, j'évoquerai la question de l'énergie. Des moyens et des innovations nucléaires doivent être redéployés.

Nous devons donc donner aux acteurs locaux les moyens législatifs raisonnables et pragmatiques, mais aussi financiers, d'agir. Sur ce volet, j'évoquerai en priorité les villes. Quelle que soit leur importance, elles sont cruciales pour l'action de la France en faveur du climat. Les mauvaises pratiques, comme l'éclairage nocturne excessif, sont à repenser. Nous devons favoriser leur transformation et permettre à chacun d'avoir un impact positif sur l'environnement. c'est aussi à chacun d'entre nous, citoyens français, qui que nous soyons, de prendre ses responsabilités individuelles et collectives, car l'action de la France- ne l'oublions pas -, c'est surtout la nôtre

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « quelle action de la France pour prendre en compte l'enjeu environnemental ? » Vaste programme, aurait dit le Général mon sens, il nous faut traduire politiquement l'urgence climatique dont parlent les scientifiques, même si le climat est un objet extrêmement complexe. Cet effort exige de nous, parlementaires, non seulement des actes concrets, mais aussi beaucoup d'humilité. Notre société est face à un défi environnemental sans précédent et notre capacité à atteindre l'objectif de neutralité carbone issu de l'accord de Paris de 2015, dont nous avons fêté récemment l'anniversaire, est remise en cause.

Je sais combien cela paraît immatériel, mais le numérique représente 10 % de la consommation électrique mondiale, soit près de 4 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Pis, ce chiffre pourrait doubler d'ici à 2025. La croissance de la pollution digitale est donc exponentielle et nos politiques publiques doivent se mobiliser pour la juguler. Aux gains environnementaux indéniables du numérique sont associés des impacts directs et quantifiables, qu'il s'agisse des émissions de gaz à effet de serre,

On a conscience de la situation, on sait quelles sont les solutions, mais il faut avoir le courage de les mettre en oeuvre. Pendant deux ans, nous avons travaillé pour élaborer un texte, désormais définitivement adopté

texte crée notamment une formation de sensibilisation à l'impact environnemental du numérique et à la sobriété numérique dans l'enseignement primaire et secondaire : c'était indispensable. Il y a un paradoxe entre l'ambition climatique des jeunes générations et leur consommation compulsive d'internet, qui engendre une grave pollution numérique. Les jeunes, comme les moins jeunes d'ailleurs, ne la comprennent pas, car ils ne la connaissent pas. Cette loi permet aussi le renforcement du délit d'obsolescence programmée et son extension à l'obsolescence logicielle, ainsi que le verdissement des centres de données, les : il s'agit Ce texte inédit constitue la première initiative législative complète sur ce sujet. Il tente d'appréhender toute la chaîne de valeur numérique, des terminaux aux centres de données en passant par les réseaux.

doivent faire évoluer leurs façons d'agir dans le secteur du numérique. En la matière, la réponse doit être européenne, claire et unanime pour que nos pays, nos entreprises, nos investisseurs et les consommateurs s'engagent sur la voie d'une transition numérique écologique.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le 21 juin 2020, après plusieurs mois de travaux, les membres de la Convention citoyenne pour le climat remettaient au Gouvernement un rapport rassemblant leurs 149 propositions pour « réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % d'ici 2030 par rapport à 1990 la Convention citoyenne pour le climat avait un objectif précis : partir des attentes des Français en matière de transition écologique pour construire des réponses adaptées. Près d'un an après la présentation du rapport, lors de l'ultime session du 28 février 2021, 96 membres de la Convention citoyenne pour le climat ont évalué les décisions du Gouvernement par rapport à leurs propositions et aux objectifs fixés. Avec une moyenne de 3,3 sur 10 pour l'ensemble des questions, le résultat est parfaitement lisible : il atteste de la grande déception des conventionnels face à l'inaction du Gouvernement. L'examen du projet de loi Climat et résilience n'a malheureusement pas permis de mettre en oeuvre les propositions ambitieuses de la Convention citoyenne Malgré un satisfecit permanent du Gouvernement, seules dix propositions des conventionnels ont été pleinement inscrites dans ce texte. Cet outil de démocratie participative était pourtant une occasion unique de traduire dans les faits les attentes et la volonté des Français sur un sujet qui nous concerne tous : la lutte contre le dérèglement climatique.

Nous l'avons constaté au cours des dernières années, avec les « gilets jaunes », qui ont fait reculer une fiscalité environnementale pourtant soutenue par une grande majorité de parlementaires, ou encore avec les nombreuses oppositions locales à des projets d'installations d'énergies renouvelables : l'acceptabilité des décisions est au coeur de cet enjeu. nous le savons -la guerre des émotions, la menace permanente ou la culpabilité ne sauraient être des solutions viables. Seule une vaste concertation démocratique, éclairée et transparente pourra ouvrir la voie à des solutions ambitieuses pour faire face au dérèglement climatique et à ses conséquences concrètes.

Alors que ce sujet anime les débats de plateau à l'approche des échéances électorales, il est consternant de voir que nos concitoyens sont mis devant le fait accompli pour des décisions stratégiques qui engagent notre avenir à tous. Tel fut le cas, par le passé,

et apportent de véritables bénéfices aux territoires. Dans mon département de la Loire, le projet d'installation d'éoliennes « Les Ailes de Taillard » en est un bel exemple. L'ensemble des collectivités territoriales concernées, les habitants des communes, les associations de protection de l'environnement et des animaux ainsi que les entreprises privées se sont rassemblés pour élaborer un projet respectueux de toutes les attentes et produisant de l'électricité pour 26 000 personnes grâce à la puissance du vent. De telles concertations permettront également de prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Ces différences, qu'elles soient météorologiques ou démographiques, météorologiques ou démographiques, doivent être prises en considération dans une logique de juste répartition des efforts entre les territoires. Il est de notre responsabilité, en tant que parlementaires, de veiller à la bonne tenue

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, dans le cadre des travaux que j'ai consacrés, en tant que rapporteur pour avis, aux crédits relatifs à la transition énergétique et au climat, j'ai pu constater les graves retards qu'accuse la France sur un certain nombre d'axes de notre politique environnementale. Pour ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, ce retard est particulièrement criant. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de voir notre pays en queue de peloton européen, d'autant plus que le dernier rapport de Réseau de transport d'électricité (RTE) montre que nous aurons nécessairement besoin d'importantes sources d'énergies renouvelables, même en relançant notre programme nucléaire.

la chaleur : il semble essentiel d'accroître largement les moyens du fonds Chaleur dès 2022. Cette piste est-elle envisagée par le Gouvernement ? En matière de lutte contre la pollution de l'air, nous ne sommes pas non plus à la hauteur. Je ne reviens pas en détail sur les diverses procédures contentieuses engagées contre notre pays-

ces structures sont touchées par la baisse tendancielle des contributions des entreprises et, parfois, par le désengagement des collectivités territoriales. Cet état de fait peut nuire à leur indépendance.

tout en maintenant leur autonomie ? En outre, j'estime que nous ne sommes pas à la hauteur en matière de gouvernance de la transition énergétique et climatique. Les moyens confiés au Haut Conseil pour le climat demeurent insuffisants, en dépit de la légère augmentation de crédits prévue par le projet de loi de finances pour 2022. Le recours à un cabinet de conseil privé pour analyser le projet de loi Climat et résilience, en début d'année, est tout bonnement scandaleux. Non seulement on peut douter de l'indépendance de l'étude réalisée, mais surtout cette mission aurait dû être confiée au Haut Conseil pour le climat, précisément créé à cette fin par le Président de la République. Sénat réclame aussi que les régions et les intercommunalités soient mieux accompagnées dans la transition, par un fléchage d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). nous oppose un refus catégorique. Comment peut-on espérer mener des politiques écologiques territorialisées sans mettre en face le financement adéquat ? Ces écarts entre le verbe et l'action, entre le « » et l'incapacité à respecter nos propres engagements climatiques, affaiblissent la voix de la France sur la scène internationale. C'est fort dommage,

au cours de ce quinquennat, que je vais vous détailler. Nous avons franchi un cap en inscrivant l'enjeu écologique dans l'ensemble de nos politiques publiques comme dans le quotidien de nos concitoyens.

nous allons plus loin encore avec le plan d'investissement France 2030, qui est largement dédié aux enjeux environnementaux. À ce titre, 8 milliards d'euros sont fléchés vers le secteur de l'énergie, notamment pour développer la filière de l'hydrogène vert et décarboner notre industrie,

en matière de justice environnementale, notamment la création du délit de mise en danger de l'environnement et, pour les atteintes plus graves, la création du délit d'écocide. Nous avons également renforcé l'échelle des peines.

des chantiers prioritaires, vous le savez, sera de renforcer le marché carbone européen, essentiel pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous voulons également avancer sur le verdissement des transports. Au début de ce quinquennat, la France a été l'un des premiers pays au monde à fixer une date pour la fin des ventes de véhicules thermiques,

Dans ce cadre, l'adoption d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est fondamentale pour éviter les risques de fuite carbone et pour que la protection de l'environnement soit un atout et une opportunité tant pour nos industries que pour les travailleurs européens.

Madame la secrétaire d'État, je concentrerai mon propos sur la prévention des risques naturels majeurs. Jeudi dernier, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est déplacée dans les Alpes-Maritimes, précisément dans la vallée de la Roya, afin de mesurer l'ampleur des dégâts et des travaux de reconstruction un un an après le passage de la tempête Alex. Onze ans après la tempête Xynthia qui a meurtri la côte Atlantique, cet événement climatique de la Roya ne sera plus un cas isolé dans les années à venir- hélas, pourrait-on dire. Hier encore, des inondations ont frappé le Nord-Pas-de-Calais. Il n'est pas exagéré de dire que les catastrophes naturelles sont devenues notre lot quotidien. Chaque année, depuis sept ans, inlassablement, j'ai alerté les gouvernements successifs sur les besoins d'accompagnement de nos concitoyens dans ces situations, tant pour la prévention des risques que pour leur indemnisation. Hélas, le fonds Barnier a plafonné, donc amputé de financements pourtant nécessaires. En 2022, il sera intégré directement au budget. Alors que la réserve de 700 millions d'euros et les 230 millions d'euros de recettes annuelles devraient être consacrés intégralement à ces actions, ce ne sera donc pas le cas l'année Pour la tempête Alex, comme Dominique Estrosi Sassone l'a indiqué ce matin lors de la séance de questions orales, certaines dépenses ne sont prises en charge ni par les assurances, ni par le fonds Barnier, ni par la dotation de solidarité.

pourrait augmenter de plus de 50 %. C'est dire l'urgence de la situation ! Le fonds Barnier, qui intervient pour aider financièrement les collectivités et mettre en sécurité les personnes exposées à ces menaces graves, devait être renforcé. Il l'a été, puisque nous pouvons observer une augmentation de 70 % du montant des crédits de ce fonds par rapport au début du quinquennat. Il a été porté à 235

L'enveloppe de la dotation de soutien à l'investissement local n'y suffira pas. Les plans et les schémas risquent de rester largement lettre morte. Depuis 2017, le Sénat adopte systématiquement la disposition relative à la dotation climat aux collectivités territoriales dans les projets de loi de finances

Alors que Bercy refuse d'avancer sur ce point, la Commission européenne semble, quant à elle, saisir l'enjeu de la dotation climat, puisqu'elle propose de flécher 100 % des recettes des ETS,,

d'avancer clairement en faveur de cette dotation aux collectivités que les réseaux climats et les territoires ainsi que le Sénat vous demandent et que les défis climatiques et environnementaux exigent sérieusement

À l'issue d'un quinquennat qui devait nous placer sur cette voie vertueuse, l'heure du bilan carbone a sonné. Lors de l'examen du projet de loi Climat et résilience, le Gouvernement a demandé au Boston Consulting Group une étude évaluant l'impact carbone de l'ensemble des mesures prises depuis 2017.

effet de serre, notamment le BTP, qui représente 27 % des émissions dans notre pays. Après des années de stagnation en matière de rénovation énergétique, le succès récent de MaPrimeRénov'est bienvenu : 700 000 dossiers devraient ainsi être validés d'ici à la fin de cette année. Ces résultats prouvent que la transformation du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) en prime d'État était très pertinente. Le caractère incitatif du dispositif a été renforcé grâce à l'extension des critères d'attribution, à compter du 1 janvier 2021, à tous les propriétaires sans condition de revenus, ainsi qu'aux copropriétés.

Il s'agit là d'une tendance lourde depuis le début de ce quinquennat et vous n'arrivez manifestement pas à stopper l'hémorragie de l'expertise publique environnementale. Le recours à des cabinets privés, tels que le Boston Consulting Group, en est l'un des exemples les plus frappants.

La séance est suspendue. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème : « La perte de puissance économique de la France- notamment en termes de compétitivité, d'innovation et de recherche -et ses conséquences sur la situation sociale et le pouvoir d'achat.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la puissance est la capacité d'un acteur à imposer ses choix aux autres acteurs- voilà un vocabulaire qui rime avec compétitivité et guerre économique. La puissance ainsi définie s'est toujours déclinée en termes de croissance. Le thème de ce débat souligne donc encore un peu plus, s'il le fallait, votre croyance sans faille, à l'instar de l'immense majorité de la classe dirigeante, dans une croissance infinie.

que notre avenir énergétique soit fossile, nucléaire ou renouvelable, le coût de l'énergie ne reviendra jamais au niveau ayant favorisé les grandes heures de la croissance. Le réalisme implique d'apprendre à vivre sans cette croissance du PIB, incompatible avec l'indispensable sobriété énergétique. Il s'agit d'un impératif vital.

Ce système économique productif, qui dépend de l'extraction et de la transformation des ressources, ne peut croître indéfiniment. Depuis les années 1980, la croissance ne permet pas non plus de réduire les inégalités en Europe et aux États-Unis ; pire, elle contribue à les creuser, ses fruits étant captés depuis quarante ans par le décile le plus riche. Heureusement, Heureusement, il me semble possible de concevoir, de débattre et de mettre en oeuvre une transformation de notre organisation et de notre économie sans miser sur le pari périlleux de la croissance.

La fiscalité demeure l'un des leviers essentiels, en France et à l'échelon européen, pour réduire les inégalités : supprimer les niches qui profitent aux plus aisés, augmenter la progressivité des impôts pour lisser les écarts de revenus ou encore imposer plus fortement le capital et le patrimoine.

le mythe d'un retour à une puissance économique forcément prédatrice n'est ni souhaitable ni même réaliste. Nous devons passer le cap de cette ère industrielle, responsable de la destruction du climat et de nos ressources, pour nous engager enfin vers une économie économe,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis trente ans, les gouvernements libéraux ont réduit les cotisations sociales et la fiscalité des entreprises pour garantir la compétitivité de l'emploi dans notre pays.

Les grandes entreprises continuent de délocaliser leur activité en Europe de l'Est et en Asie. Les dividendes des actionnaires ont explosé et les salaires ont stagné. Alors que le niveau de chômage n'a jamais été aussi élevé et que l'emploi industriel est en baisse depuis 2019, Emmanuel Macron a annoncé un nouveau durcissement des critères de l'assurance chômage, qui s'ajoute à la réforme de septembre

il réduit les droits sociaux et rechigne à compenser l'augmentation du prix de l'énergie pour tous nos concitoyens. Nous, parlementaires communistes, défendons un projet radicalement opposé, qui vise à qui vise à permettre à chacun de vivre dignement de son travail, aux jeunes d'accéder à des emplois stables, aux populations de disposer partout de services publics de qualité, au pays de se doter de nouveau d'une industrie à la fois garante de notre souveraineté répondre aux besoins de la société. Pour y parvenir, il nous faut réorienter radicalement les richesses vers la satisfaction des besoins des femmes, des hommes et des jeunes, plutôt que de toujours engraisser les plus riches et les marchés financiers, et confier de vrais pouvoirs de décision aux citoyens et au monde du travail. Emmanuel Macron a multiplié les cadeaux fiscaux à une poignée d'ultra-riches et au capital : 358 000 familles, dont le patrimoine

le travail crée des richesses. Face aux libéraux et aux tenants de l'austérité budgétaire, nous voulons une économie au service de l'humain. De 2008 à 2017, l'Union européenne a apporté 1 500 milliards d'euros au système financier, ait modifié la courbe du chômage. À l'inverse de ceux qui invoquent le défaitisme et la défaite morale de la France, nous prônons les jours heureux. Nous proposons une autre utilisation de l'argent pour produire autrement et partager les richesses. Pour que chacun puisse vivre dignement, il faut augmenter les salaires. Pour donner du travail au plus grand nombre, il faut réduire le temps de travail hebdomadaire à 32 heures et recruter massivement dans la fonction publique. Mais bien sûr ! Nous avons besoin de développer les services publics, d'investir dans la santé et en faveur d'une autre industrie. Face à l'urgence sociale, nous devons augmenter le SMIC de 200 euros net par mois, revaloriser les pensions et les minima sociaux, appliquer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,

Face à l'urgence sociale, il faut aussi baisser le prix des carburants et réduire de 30 % les taxes sur le gaz et l'électricité. Le déclin de la puissance économique de la France est la conséquence des choix budgétaires des gouvernements successifs. Il est encore temps d'inverser la tendance en adoptant une politique orientée vers l'investissement et l'humain plutôt que vers l'austérité et le marché. Vive l'austérité

monsieur le ministre, mes chers collègues, les inquiétudes quant à la dégradation de la compétitivité du tissu productif français sont bel et bien fondées. la covid-19, la crise économique et la désorganisation des chaînes de production ont touché tous les pays européens en 2020, la France semble avoir particulièrement souffert.

Si l'on inclut les services, le constat est malheureusement le même : les exportations de biens et de services de la zone euro ont reculé de 13,2 % l'an passé, tandis que celles de la France ont littéralement plongé de 19,3 %.

expliquer la contre-performance française. L'Italie et l'Espagne ont pris des mesures de distanciation sociale plus strictes que nous sans avoir enregistré de pertes de parts de marché. Cela laisse donc supposer une fragilité générale de l'appareil productif français en 2020. Certains économistes craignent que notre pays soit confronté à une nouvelle phase de désindustrialisation dans les prochaines années, alors même que le Gouvernement investit massivement dans un plan de relance de 30 milliards d'euros, largement relayé par les préfets dans nos territoires.

trop compliqué », « encore un plan de plus », « trop d'objectifs confus, « 2030, c'est loin » ... Comment expliquez-vous, monsieur le ministre, le peu d'engouement des acteurs économiques, à quelques exceptions Au-delà du plan de relance, quelles solutions s'offrent aujourd'hui à la France pour renouer avec la compétitivité et le pouvoir d'achat ? Avec un déficit public important, un déficit extérieur qui se creuse et des dépenses publiques très élevées, la France est un pays atypique au sein de la zone euro. Quel nouveau modèle de croissance durable devons-nous privilégier si nous voulons éviter tout ajustement brutal des salaires et des dépenses publiques qui pourrait se dessiner après l'élection présidentielle ?

critères environnementaux coûteux qui affectent la productivité de nos agriculteurs, n'orchestre-t-elle pas, finalement, une nouvelle perte de compétitivité agricole de l'Europe ? Ne va-t-elle pas à rebours des priorités de pouvoir d'achat de nos concitoyens et de la nécessité de nourrir la planète ?

Le présent débat aurait alors trouvé toute sa place dans cette discussion et aurait pu se traduire en propositions d'amendements. Le déclin économique de la France et ses inévitables conséquences sociales, dont le mouvement des gilets jaunes est l'exemple le plus prégnant de cette législature, est un vaste sujet.

2010 en Europe et de l'émergence de nouveaux acteurs extra-européens, au premier rang desquels la Chine. Il s'agit donc d'abord d'une perte de puissance relative. Nous sommes confrontés à l'affirmation d'autres puissances poursuite du leadership technologique des États-Unis en ce début de XXI siècle, dans des domaines comme le numérique, le spatial, les biotechnologies ; réaffirmation de la puissance allemande au coeur de l'Europe à la suite du grand élargissement de l'Union européenne vers l'Est surtout, émergence spectaculaire de la Chine depuis deux décennies après son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avec la construction de monopoles de fait dans la production de certains biens ou matériaux comme les terres rares. D'autres pays et régions du monde émergent en Asie, en Amérique latine au Moyen-Orient. Nous assistons à une « désoccidentalisation » du monde comme conséquence ultime de la mondialisation, pour prendre le contrepied de l'expression de l'économiste Serge Latouche.

Cette croissance, dite « fondée sur la consommation », se paye aujourd'hui comptant avec le renchérissement de produits énergétiques ou des matériaux de base, comme dans la construction, et un impact direct sur le pouvoir d'achat. Le bouleversement économique lié à la pandémie n'a pas modifié cette réalité, alors que le déficit commercial s'est encore élevé à plus de 60 milliards d'euros en 2020. À l'inverse, la reprise de cette année et l'inflation qui s'ensuit révèlent les faiblesses de notre appareil productif et notre dépendance à l'extérieur. Cela fait des années que certains experts ou responsables alertent sur la dégradation de la position économique de la France. Des efforts pour réhabiliter la production française auprès des consommateurs ont certes été réalisés pense, par exemple, au salon du, qui s'est tenu voilà quelques jours à la porte de Versailles. Il faut reconnaître le caractère précurseur des idées défendues en son temps par l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg. aujourd'hui combien notre dépendance se paye cher. Il nous faut retrouver notre souveraineté industrielle, alimentaire, pharmaceutique, même si cela doit coûter un peu plus cher. Dans le même temps, il faut augmenter les salaires les plus bas et revoir la réglementation des marchés publics. marchés publics. La seule loi de l'offre et de la demande n'apporte pas de réponse satisfaisante dans bien des domaines comme la santé, l'éducation ou encore l'agriculture. Il faut en profiter pour mettre en place à nos frontières des taxes carbone, afin de rééquilibrer nos échanges internationaux, ainsi que des exigences en matière de normes sociales et environnementales, ce que certains ont pu appeler le « juste échange Enfin, nous avons intérêt à davantage produire chez nous, ou près de chez nous, afin de nous prémunir du risque géopolitique et contribuer à la réindustrialisation de nos territoires et au développement des pays les plus proches, comme, par exemple, ceux du Maghreb. que la France et l'Europe réinvestissent massivement dans les secteurs d'avenir. Est-il toujours acceptable et sûr que la plupart de nos microprocesseurs proviennent de Taïwan ou encore que nos médicaments soient de plus en plus fabriqués en Inde Pour cela, il faut aussi réinvestir massivement dans la recherche publique, trop délaissée au cours des dernières années. Si nous ne travaillons pas ensemble sur ces enjeux, notre positionnement sur l'échiquier international va nous échapper.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans son discours de réception du prix Nobel de littérature, Albert Camus disait Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Pour des raisons différentes de celles de 1957, cette phrase garde, pour les générations d'aujourd'hui, toute sa force d'appel au devoir et à la responsabilité. Je crois que l'on ne peut débattre utilement de la puissance économique de la France sans se poser la question de la place qui doit être la sienne dans la fin de la « civilisation du carbone » et ses conséquences. C'est d'abord d'une trajectoire de transition de modèle, comprise par le plus grand nombre, dont nous avons urgemment besoin. La France ne peut ignorer « l'apparition ou l'irruption du terrestre dans notre Histoire », pour reprendre la belle idée de Bruno Latour. Aujourd'hui, sous le triple effet de la réception des thèses écologistes dans l'opinion, des démarches scientifiques prédictives et des effets dévastateurs et bien concrets des pollutions et du réchauffement climatique, les prises de conscience progressent. Mais, au-delà des paroles, peu sont ceux qui donnent un contenu au projet global de transformation du système productif. De COP en COP, les constats désabusés se succèdent. Pour autant, il serait injuste d'oublier ou de dénigrer les changements de stratégie engagés dans nombre d'entreprises françaises des secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'agriculture, de l'énergie ou du recyclage, par exemple. de « transition-coopération-compétition » qui a débuté entre les économies du monde, la France doit définir très rapidement sa stratégie. de justice sociale, elle doit transformer souverainement ses politiques pour être plus attractive, pourvoyeuse d'emplois utiles et bénéfiques à l'écoumène. L'éducation générale et populaire, l'enseignement supérieur et la recherche, l'accueil des étudiants étrangers, la souveraineté numérique, la formation générale et professionnelle tout au long de la vie, la culture font partie de ces domaines ou processus qui feront le monde de demain et notre place dans le monde de demain.

Dans ce contexte d'urgence, l'avenir économique de la France, sa compétitivité, ses emplois, son modèle social et culturel passeront par sa capacité à changer de référentiel dans de nombreux domaines.

Sur le plan de la gouvernance et des institutions, il rappelle que transformer la richesse comptable en biens institutionnels et symboliques et constituer un patrimoine social pour l'ensemble de la société est la tâche que se fixe le régime républicain. La République est un dispositif d'accumulation du patrimoine matériel et symbolique pour lequel l'ensemble de la communauté s'organise, en république précisément, pour mieux le gérer et en assurer sa conservation. La notion de richesse doit être réinterrogée, une des tâches du politique étant de transformer les richesses matérielles et financières en biens juridiques, sociaux, culturels et symboliques. Aujourd'hui, on pioche dans le patrimoine institutionnel et social en précarisant les statuts, en fragilisant le droit du travail et en réduisant la protection sociale. « Et dans les conditions actuelles, la croissance passe nécessairement par la désinstitutionalisation des sociétés à l'accélération de laquelle s'attache la gouvernance, avatar néolibéral du gouvernement des hommes. « Or il n'y a pas de développement durable possible sans le renforcement du processus de patrimonialisation institutionnelle, sociale et symbolique. À travers la constitution de ce patrimoine, nos activités témoignent de leur capacité à construire de la durée. « Et aucun membre de la communauté nationale, quel que soit son statut, ne doit être écarté de la construction de cette " durée

La responsabilité doit s'imposer comme la « colonne vertébrale de l'éthique du XXI siècle ». La mise en oeuvre d'un développement vraiment durable passe aussi, et nécessairement, par la transformation de la responsabilité pour répondre aux défis actuels. C'est donc au prix d'une reconsidération du politique et de l'éthique que les générations actuelles et futures éviteront « que le monde se défasse » et que l'économie française

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux entamer ce débat en partageant avec vous une conviction : il n'y a pas de souveraineté nationale sans puissance économique.

voire de « déclinisme »- nous nous y refusons ! Bien sûr, nous avons tous à l'esprit certains exemples qui nous invitent à établir un diagnostic assez sombre de la situation. situation. Notre incapacité à produire un vaccin contre la covid, par exemple, a été un traumatisme au pays de Pasteur. Toutefois, ce serait ignorer les preuves démontrant que la situation s'est améliorée au cours des dernières années. Ainsi, la France est devenue le premier pays d'Europe en matière d'investissements étrangers. Partout, dans nos territoires, des entreprises se créent qui inventent et développent les solutions de demain. Ne cédons pas à la facilité de l'autodénigrement. Pour apprécier la perte de puissance économique de la France, il faut s'en remettre à des critères objectifs, tels que le produit intérieur brut. Or, si l'on regarde l'évolution du PIB sur le temps long, deux tendances se dégagent. D'une part, la puissance économique de la France n'a cessé de croître depuis le premier choc pétrolier, à deux exceptions près la crise financière de 2008 et la crise sanitaire actuelle D'autre part, la contribution du PIB de la France au PIB mondial est passée de 6 en 1975 à 3 % en 2020. Autrement dit, si la puissance économique de la France diminue, c'est d'abord parce que la puissance économique d'autres pays, singulièrement en Asie, augmente. La perte de puissance de la France est donc relative. Relative, certes, mais aussi indéniable : si l'Occident, de manière générale, a cédé du terrain à l'Orient, la France a moins bien résisté que d'autres à ce grand bouleversement. Dans la même période de temps, le PIB du Royaume-Uni est ainsi passé de 4 % à 3 %, celui des États-Unis de 28 % à 25 %. Ces éléments de comparaison internationale démontrent une spécificité française, et pour cause : la puissance économique repose sur la compétitivité. Il ne suffit pas que le PIB croisse ; il faut qu'il croisse plus vite qu'il ne croît dans d'autres pays. Nous aurions tort d'opposer compétitivité économique et progrès social, ou même, de façon plus caricaturale, entreprises et salariés. Nous devons garder à l'esprit que la prospérité de notre économie garantit la solidité de notre modèle social. Sans compétitivité, pas de solidarité possible. Alors que des débats politiques importants nous attendent dans les prochains mois, je crois nécessaire de rappeler cette évidence : le renforcement de la compétitivité française est la clé de notre puissance économique. À cet égard, trois facteurs ont été déterminants ; ils le resteront dans les années à venir. Premièrement, il faut poursuivre la baisse des prélèvements obligatoires. Le travail mené au cours des dernières années a été remarquable, avec 50 milliards d'euros de pression fiscale en moins, dont la moitié pour les entreprises. La baisse du taux de l'impôt sur les sociétés de 33 % à 25 %, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune ou encore la baisse des impôts de production sont des mesures qui vont dans le bon sens. Elles ont restauré l'attractivité de la France. Deuxièmement, il faut bâtir un continuum d'innovation français, qui va de la recherche fondamentale au développement industriel. La réindustrialisation de la France doit investir les futurs domaines de l'excellence industrielle. À cet égard, le plan France 2030, présenté par le Président de la République, ouvre des perspectives ambitieuses. Il faut s'assurer que la recherche puisse se convertir en innovations industrielles, car c'est souvent là que le bât blesse. C'est tout l'objectif de la mission d'information que notre groupe vient de lancer, sur l'initiative de ma collègue Vanina Paoli-Gagin. Le dernier point découle logiquement des deux premiers : en améliorant la compétitivité du site France et en bâtissant les usines du futur, notre pays devra créer de l'emploi sur le territoire national à tous les niveaux de qualification afin d'améliorer, par notre outil industriel, la situation sociale et le pouvoir d'achat. Mes chers collègues, je le redis, la souveraineté nationale passe par la puissance économique. Je sais que nous sommes nombreux ici à partager cette conviction. Toutefois, pour élaborer des propositions efficaces, nous aurions tort de noircir à l'excès le tableau. L'ambition politique ne se mesure pas à la gravité du constat.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'en aborder les conséquences sociales, permettez-moi d'évoquer en premier lieu la perte de puissance économique de notre pays, fait générateur du débat qui nous est proposé aujourd'hui. Quel jugement peut-on porter sur la France en tant que puissance économique en 2021 ? Cette question renvoie inévitablement à la polémique insupportable entre des « déclinistes » à tendance masochiste et des optimistes béats, adeptes de la méthode Coué façon « argent magique »- si vous voyez ce que je veux dire. Soyons clairs le décrochage de l'économie française est malheureusement une triste réalité. Les Alstom, Pechiney, Saint-Gobain et autres Usinor, qui fleuraient bon les Trente Glorieuses, ont plutôt désormais des relents de Bérézina, Trafalgar ou Waterloo, selon que vous aurez le pied marin ou l'humeur « fantassine ... Force est de constater, pourtant, que la France n'est pas à ce jour disqualifiée à la hauteur de ce que suggèrent ses plus ardents procureurs dans leurs réquisitoires. Elle demeure en 2021, selon les analyses, la cinquième ou sixième économie mondiale au regard de son PIB. La France n'a donc pas encore quitté la cour des grands, mais elle est à deux doigts de le faire : ses dynamiques principales sont très mal orientées, ce qui est extrêmement préoccupant. L'un des pires marqueurs réside certainement dans le décrochage des parts de marché françaises à l'export voilà plus de dix ans que la balance commerciale de la France est déficitaire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation dégradée, mais la raison fondamentale réside avant tout dans la perte de compétitivité de notre pays et la faiblesse de sa stratégie à l'export. Qu'il s'agisse de spécialisation industrielle, d'orientation géographique des exportations ou de l'appareil productif, on constate une inadaptation à l'environnement, née de la globalisation économique. Longtemps, la stratégie française fut d'abandonner les productions à faible valeur ajoutée et intensives en main-d'oeuvre peu qualifiée pour se spécialiser dans les industries du savoir à forte valeur ajoutée. L'un des postulats sous-jacents à cette stratégie était que les pays émergents, auxquels étaient laissées les activités à faible valeur ajoutée, resteraient cantonnés à ce rôle, dans un contexte d'entrée dans un monde post-industriel où la France pourrait faire preuve de son « génie » national et ainsi créer de la valeur. C'était la mondialisation heureuse, les nouveaux marchés, les nouveaux débouchés, dont la et les premiers de cordée sont les derniers avatars. La réalité est tout autre, avec des répercussions sociales particulièrement brutales. La part de l'industrie manufacturière dans l'économie française a diminué de moitié, passant de 22,3 % à 11,2 %, et représente 3,1 millions d'emplois directs en France,

Deux autres conséquences majeures sont la montée du séparatisme social et l'affaiblissement de la démocratie, au moment même où notre pays devrait être rassemblé pour affronter efficacement les multiples crises auxquelles il est confronté. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une nation très ouverte à l'économie mondiale ne puisse être une démocratie moderne. Loin de là. L'État-nation doit être en capacité de maîtriser l'intensité de son ouverture économique pour ne pas nuire à ses compromis démocratiques et sociaux fondamentaux. La mondialisation libérale et la libération de la finance ont profondément déréglé les équilibres planétaires. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement temporaire. Le capitalisme coexiste de plus en plus difficilement avec les nations démocratiques, ces communautés humaines pluriséculaires liées par une langue ou une histoire communes, et plus encore par la volonté de se gouverner elles-mêmes. Par ailleurs, l'environnement administratif, légal, fiscal et social entrave la montée en puissance de la compétitivité française, sur laquelle pèsent trop de contraintes. Les approches comptable et bureaucratique à courte vue sont aussi mortifères que le capitalisme de la rente. La France dispose pourtant d'immenses atouts. Plutôt que d'opposer systématiquement secteurs public et privé, il est grand temps de comprendre que c'est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés qui sont devant nous.

Je ne peux que partager une telle position. L'économiste rappelle la nécessité d'un meilleur financement de notre recherche fondamentale. C'est

comme je le rappelle dans mon rapport pour avis, initialement budgétaire, et transformé en rapport d'information, portant sur les crédits consacrés à la recherche, à l'enseignement supérieur et au spatial, les deux tiers de la recherche en France sont le fruit de l'investissement des entreprises. je ne peux que regretter la suppression du doublement du crédit d'impôt recherche (CIR) destiné aux entreprises qui collaborent avec des organismes de recherche et déplorer la baisse de créances anticipée de 161 millions d'euros. La recherche doit se tourner vers les innovations de rupture, par exemple dans les domaines de l'énergie, de la santé, du spatial ou de l'alimentation. Or de telles innovations impliquent un passage- difficile -de la recherche fondamentale au champ des applications. des applications. La recherche partenariale est indispensable entre opérateurs publics et entreprises privées, en ce qu'elle permet de sécuriser des briques technologiques et de favoriser les transferts des acquis de la recherche fondamentale vers l'innovation et les applications industrielles. l'innovation n'est pas forcément verte. C'est tout l'intérêt de l'intervention étatique, qui est en mesure de diriger cette recherche vers des innovations durables. Pensons à l'hydrogène vert, qui pourrait être produit par un nouveau nucléaire, bien plus économe en déchets, et qui pourrait constituer un levier de décarbonation des industries lourdes comme la sidérurgie. C'est également en repensant la politique de la concurrence, adaptée à l'ère du digital, qu'il sera possible de relancer l'innovation, en remettant en cause des acteurs devenus hégémoniques qui inhibent l'innovation de leurs concurrents. Dès lors, il est impératif d'arriver à rapatrier une partie de la production industrielle délocalisée. Il faut casser le cercle vicieux qui consiste à réduire nos émissions nationales par la désindustrialisation, tout en augmentant de 50 % nos émissions importées. Je pense notamment, dans mon département de Lot-et-Garonne, à l'industrie pharmaceutique. Je salue ainsi la présentation du plan France 2030, qui agit sur les innovations de rupture tout en rappelant la nécessité d'assurer un cadre pérenne de financement de la recherche. je salue les objectifs de sécurisation de l'accès aux matériaux stratégiques tels que les terres rares, ainsi que la circularité accrue de la production au recyclage - je pense, notamment, aux indispensables batteries. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, système social obsolète, incapacité à mener des réformes, système d'innovation médiocre, dégradation de la compétitivité : ce tableau du décrochage de l'économie française est un point de vue. Force est de constater que l'économie française n'est pas, à ce jour, disqualifiée à la hauteur de ce qui est suggéré par ses détracteurs. En termes de PIB, la France est toujours la sixième puissance mondiale. Elle demeure aussi le cinquième exportateur de biens et services. Est-ce à dire que la situation sociale est bonne et que le pouvoir d'achat des Français progresse ? La période du covid-19 a démontré la capacité du pays à protéger son économie et à maintenir un niveau de revenus grâce au chômage partiel et au soutien inconditionnel des entreprises, certes rendu possible par le « quoi qu'il en coûte. Le visage de notre industrie a beaucoup changé avec les nouvelles technologies de l'information. Certains secteurs se renforcent, comme l'industrie agroalimentaire, premier employeur industriel du pays, qui contribue fortement à la dynamique de l'emploi. Malheureusement, la crise du covid-19 a révélé notre haut niveau de dépendance sur des produits déterminants pour notre activité et notre sécurité. Malgré la crise sanitaire, le pouvoir d'achat des Français aurait augmenté, selon chiffre cache une autre réalité et de grandes disparités. Certains de nos concitoyens sont davantage exposés à la pauvreté : chômeurs, familles monoparentales, jeunes, retraités La contrainte de plus en plus forte sur le budget des ménages les plus modestes est une hausse continue des dépenses dites préengagées : loyers, remboursement d'emprunt, abonnements, assurances ... Selon France Stratégie, ces dépenses sont passées de 27 % de la dépense totale des ménages en 2001 à 32 % en 2017. En cette fin 2021, ces dépenses contraintes augmentent avec les prix de l'énergie : hausse de 16 % pour l'essence, de 6,3 % pour l'électricité, de 19,5 % pour les loyers. Les prix de l'alimentation flambent également.

On observe également un rebond du travail indépendant, de l'ubérisation, avec une protection sociale lacunaire et une augmentation du nombre de travailleurs à faibles revenus. Les inégalités se creusent en France : depuis 2018, les riches sont devenus plus riches, et les pauvres plus pauvres et plus précaires, faisant le yo-yo entre emploi et chômage. Le ruissellement attendu n'a pas eu lieu. La baisse des allocations logement, la réforme de la fiscalité du capital et, désormais, la réforme de l'assurance chômage, contribuent à l'augmentation des écarts de niveau de vie entre Français. La première parade pour lutter contre ces inégalités est de garantir au travailleur une juste rémunération, qui lui permette de vivre dignement, sans privation majeure. En 2019, 19 % des Français se percevaient comme pauvres contre 13 % en 2017. La mutation industrielle doit se traduire par l'émergence d'une industrie tournée vers la transformation de notre société, au service du progrès social et écologique. Un plan de relance mieux ciblé sur les secteurs stratégiques eût été une belle opportunité, que votre Gouvernement n'a pas saisie. Ce n'est que grâce aux transferts sociaux et fiscaux que le niveau de vie global a pu se maintenir. Cela se traduit par une forte augmentation du nombre des bénéficiaires de minima sociaux, en hausse de 30 % depuis 2008, ce qui a suscité un sentiment de déclassement chez une partie des Français. Le système de redistribution protège, mais chacun aspire plutôt à recevoir une juste et digne rémunération de son travail. Notre pays dispose de la richesse suffisante pour permettre à nos concitoyennes et concitoyens de disposer des ressources nécessaires pour vivre dignement, grâce à une meilleure répartition des richesses.

70 % de l'érosion de l'excédent agricole s'expliquent par un effet de compétitivité négative, entraînant une augmentation des importations.

Déclin ou déclassement ? Oui, la France perd du terrain. Le taux de pauvreté, passé de 13,6 % en 2009 à 14,8 % aujourd'hui, en témoigne. Politique familiale, éducation, formation, innovation, réindustrialisation doivent être les champs de reconquête, dans un contexte européen privilégié. Le frein majeur reste un État trop lourd, bureaucratique, qui retarde les projets et ne laisse pas assez de liberté aux chercheurs, aux entrepreneurs et aux territoires. Combien de projets ont échoué, comme nous pouvons le voir dans les Hauts-de-France, monsieur le ministre, face à la concurrence d'un pays voisin comme la Belgique, plus ouverte conditions d'installation, ou à celle du Canada et des États-Unis pour nos jeunes chercheurs ? La richesse ne ruisselle ni sur les ménages ni sur les territoires ; source d'inégalités, elle génère un sentiment d'appauvrissement et d'abandon. Elle doit trouver une plus juste répartition avant et après production : avant, par la formation ; après, par une meilleure rémunération du travail, plutôt que de reposer sur un système social à bout de souffle, parmi les plus redistributifs, au prix d'un endettement massif et d'un poids des prélèvements obligatoires toujours plus élevé, à 47,4 % du PIB, soit le plus haut de l'Union européenne. Pour reconquérir souveraineté et grandeur, comment accélérer notre croissance, assurer une répartition équitable de la richesse induite et rétablir en même temps les comptes de la Nation ? le ministre déclarait : « La France est droguée à la dépense publique. » Au-delà de la crise, qui a redonné corps à l'Union européenne, et au-delà de la solidarité de la BCE, on attend des actes tangibles de convergence réglementaire, sociale, fiscale,

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre de la perte de puissance économique de la France et ses conséquences sur la situation sociale et le pouvoir d'achat. Plutôt que d'une France en perte de vitesse, permettez-moi de parler aujourd'hui d'une France devenue, depuis 2019, le pays le plus attractif en Europe d'une France qui, à la sortie de la crise économique, enregistre le rebond le plus fort ; d'une France qui retrouve sa place parmi les économies les plus dynamiques en Europe. Mesdames, messieurs les sénateurs, c'est un constat : ces dernières décennies ont été marquées par une perte de compétitivité, par une désindustrialisation, par la destruction de l'appareil productif et par un chômage de masse. les dynamiques constatées depuis 2017 montrent que cette situation n'est pas une fatalité. Elles ont prouvé qu'une politique publique volontariste peut venir démentir ceux qui se complaisent dans le déclinisme. La France a connu depuis 2017 une croissance plus importante que ses principaux partenaires européens. La compétitivité française s'est redressée, avec des coûts salariaux unitaires maîtrisés grâce aux baisses d'impôts et de charges mises en oeuvre par le Gouvernement. Je pense à la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, qui passera de 33,3 % à 25 % d'ici à 2022, se rapprochant ainsi du taux moyen de la zone euro. Je pense aussi à l'allégement pérenne des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Je pense enfin à la baisse des impôts de production, qui pèsent sur l'investissement des entreprises, en particulier dans l'industrie, d'un montant pérenne de 10 milliards d'euros à partir de 2021.

Ce dynamisme sur le marché de l'emploi se poursuit en sortie de crise sanitaire grâce à la protection inédite des entreprises et des salariés que nous avons mise en place. Le taux de chômage n'a pas augmenté. Il y a plus d'emplois aujourd'hui qu'avant la crise. Au total, un million d'emplois ont été créés depuis 2017. Pendant le quinquennat, le dynamisme s'est accompagné d'une amélioration de la qualité de l'emploi, avec une augmentation de la part des CDI et une baisse des temps partiels. Le taux d'emploi en CDI des personnes âgées de 15 à 64 ans a augmenté de 1,3 point entre 2017 et 2021. Pour permettre l'accès du plus grand nombre à un emploi tout en améliorant l'efficacité du marché du travail, le droit du travail a été simplifié. Les ordonnances de 2017 tendent à offrir plus d'égalité, de liberté et de sécurité, aux salariés comme aux entrepreneurs, en renforçant le dialogue social. Pour faciliter la montée en compétence de tous les actifs, le système de formation professionnelle a été rénové et renforcé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui réforme la formation continue et l'apprentissage. Un effort tout particulier a été déployé en faveur du développement des compétences par la mobilisation de 15 milliards d'euros dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Fin 2020, plus d'un million de personnes éloignées de l'emploi ont déjà été formées. les dispositifs de formation ont été renforcés par le plan France Relance, à autour de 3 milliards d'euros, le dispositif Pro-A, qui vise à favoriser le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés par une formation en alternance, et le dispositif Transitions collectives, qui repose sur une mise en relation de l'offre et de la demande de compétences à l'échelon local. Les mesures en faveur de l'apprentissage donnent déjà des résultats exceptionnels. Nous sommes en train de gagner cette bataille de l'apprentissage, avec plus de 500 000 apprentis en 2021, alors que nous en comptions moins de 280 000 en 2016. Le redémarrage rapide de l'économie, à la sortie de la crise, a créé des tensions sur le marché de l'emploi, avec des difficultés de recrutement du côté des entreprises. Le plan de réduction des tensions de recrutement, dont l'enveloppe s'élève à 1,4 milliard d'euros pour 2021 et 2022, vise à pallier ces limites. limites. Alors que les entreprises font face à une pénurie de main-d'oeuvre, la réforme de l'assurance chômage, qui sera finalisée d'ici à la fin de l'année, viendra compléter l'action du Gouvernement en faveur de l'emploi. L'amélioration de la compétitivité de nos entreprises passe également par les investissements dans l'innovation et dans la recherche et développement. L'investissement dans l'innovation a été et demeure une priorité. Au-delà de la reconduction des aides fiscales en faveur de l'innovation- je pense au crédit d'impôt recherche (CIR) et au régime des jeunes entreprises innovantes ou crédit d'impôt innovation -, nous avons lancé, au mois de janvier 2021, la quatrième vague du programme d'investissements d'avenir (PIA4), d'un montant de 20 milliards d'euros. Cette nouvelle édition du PIA va notamment permettre de financer les stratégies d'accélération et l'innovation de rupture, avec des objectifs technologiques précis et ambitieux. La compétitivité de nos entreprises passera enfin par les nécessaires transformations numériques et écologiques. Nous investissons pour accompagner les entreprises françaises avec le plan France avec le plan France Relance, qui consacre 30 milliards d'euros aux enjeux de la transition écologique et soutient massivement la numérisation et la modernisation de l'appareil productif des PME. Le plan d'investissement France 2030 complète et prolonge l'action du Gouvernement pour la reconquête industrielle en soutenant l'émergence de nouveaux champions innovants dans des secteurs porteurs. Ce plan, doté de 34 milliards d'euros, répond aux grands défis de notre temps, en particulier la transition écologique, à laquelle la moitié des crédits seront consacrés. Il cible dix filières stratégiques dans lesquelles nous avons l'ambition de faire émerger les futurs champions technologiques de demain. Il s'agit d'accompagner la transformation de nos secteurs d'excellence.

Le projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, que j'ai eu la chance de présenter devant le Sénat voilà quelques semaines, s'inscrit dans la continuité de ces textes. Au-delà de ces mesures transversales, le Gouvernement a mis la réindustrialisation de notre économie au coeur de son action, puisque l'industrie est indispensable pour notre souveraineté, pour la résilience de notre économie et pour la vitalité de nos territoires. Ainsi, 35 milliards d'euros sont aujourd'hui mobilisés en faveur de l'industrie dans le cadre de France Relance. secteur est aussi au coeur du plan France 2030. Ce choix s'appuie sur une conviction profonde : celle de la nécessité d'avoir un secteur productif fort pour faire face aux défis de la mondialisation et aux transitions du monde de demain. Vous le voyez, depuis 2017, le Gouvernement n'a eu de cesse d'oeuvrer pour améliorer la compétitivité et la résilience de notre économie et pour remettre la France sur les rails d'une croissance forte et durable. Mesdames, messieurs les sénateurs, la politique économique ambitieuse du Gouvernement s'est accompagnée d'une action forte en faveur du pouvoir d'achat des Français et de la lutte pour l'égalité des chances. Pour que le travail paye mieux et soit rémunéré à sa juste valeur, le Gouvernement a pris plusieurs mesures visant à diminuer les prélèvements qui pèsent sur le travail, à encourager l'activité et à soutenir le pouvoir d'achat. La revalorisation de la prime d'activité de 100 euros au niveau du SMIC, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macron, qui peut être versée jusqu'au début de la réduction de l'impôt sur le revenu des classes moyennes, l'exonération des heures supplémentaires de cotisations salariales et d'impôt sur le revenu, ainsi que les mesures en faveur du développement de l'intéressement et de la participation permettent que le travail paye mieux. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour tous les contribuables complète ces mesures de justice et de pouvoir d'achat. Pour lutter contre les inégalités de destin, des dispositifs se concentrant sur l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi ont été renforcés, notamment pour les jeunes, avec le plan « 1 jeune, 1 solution » et la mise en place dans les prochains mois du contrat d'engagement jeune. Des mesures importantes ont également été mises en oeuvre pour soutenir les plus vulnérables dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, avec la revalorisation de minima sociaux ou la réforme 100 % santé. Le soutien aux plus précaires a été un axe fort de la gestion de la crise, avec la prolongation des revenus de remplacement, tels que le revenu de solidarité active (RSA), et le versement d'allocations exceptionnelles. Il s'est prolongé au sein de France Relance avec la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire et le soutien aux aux associations luttant contre la pauvreté. Par ailleurs, pour protéger les Français face à la hausse des prix, une indemnité inflation de 100 euros sera versée en fin d'année et en début d'année prochaine à environ 38 millions de Français, dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros net par mois. Les prix du gaz seront gelés à partir du mois d'octobre, et ce jusqu'à la fin de l'année 2022. La hausse des tarifs réglementés de l'électricité sera limitée à 4 % au mois de février 2022, le levier de la fiscalité, contre une hausse initialement attendue de plus de 15,7 15,7 % à cet horizon. En définitive, le pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages a progressé de manière continue depuis 2017, de 8 % en moyenne sur le quinquennat. Les Français, à tous les niveaux de revenus, ont bénéficié des mesures fiscales et sociales du quinquennat. Ceux qui ont le plus gagné, ce sont les Français qui travaillent et qui aspirent légitimement à vivre dignement de leur travail. Un salarié au SMIC peut ainsi gagner 170 euros de plus par mois grâce aux mesures que nous avons mises en place. Mesdames, messieurs les sénateurs, aujourd'hui, nos résultats économiques sont là : une prévision de croissance de 6,25 % pour l'année 2021 publique ! Ces résultats économiques proviennent d'abord du travail de fond que nous avons engagé depuis le début du quinquennat, mais aussi de notre stratégie du « quoi qu'il en coûte » pendant la crise, qui a permis de préserver le tissu économique. Ils proviennent enfin de notre stratégie d'investissement, avec le plan France Relance, dont le déploiement avance rapidement, et le plan France 2030, qui sera mis en oeuvre dès le début 2022.

L'Observatoire de la métallurgie pointe le risque de perdre encore 50 % des emplois d'ici à 2035. Avec la fin du moteur thermique, les secteurs des fonderies ou des composants diesel, par exemple, vont décliner rapidement. Que faire pour éviter les drames économiques et sociaux, alors que le développement de l'électromobilité ne pourra compenser entièrement le phénomène ? Il est temps de définir une voie stratégique de décarbonation du secteur tout en favorisant la création d'activités industrielles

le contrat de coalition, à accélérer et soutenir fortement la transformation de la filière automobile afin d'atteindre les objectifs climatiques tout en préservant les emplois et la valeur ajoutée. Pour limiter les pertes d'emplois, il s'agit de miser sur le développement de filières durables, d'engager des investissements importants, non seulement dans la transformation des outils de production et de distribution, mais également dans les formations et les reconversions.

Dans ce combat, l'industrie a un double rôle à jouer : d'une part, en décarbonant ses procédés ; d'autre part, en mettant au point les solutions décarbonées de demain. Afin d'atteindre notre objectif de réduction des gaz à effet de serre, l'État a mobilisé, dans le cadre de France Relance, 1,2 milliard d'euros pour soutenir et accompagner la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel. Au total, les dispositifs mis en place soutiennent d'ores et déjà 141 projets représentant 2 milliards d'euros d'investissement et 758 millions d'euros d'aides.

mais elle représente un défi sans précédent pour la filière automobile française. La transition électrique conduira nécessairement à des restructurations dans les secteurs les plus affectés. Par ailleurs, le risque de recomposition des chaînes de valeur à l'échelle mondiale, au détriment de la France et de l'Europe, existe bel et bien, menaçant nos emplois et nos savoir-faire. C'est ce qui a failli arriver dans le secteur des batteries. Les évolutions réglementaires à venir- je pense à la norme Euro 7, au paquet, avec l'arrêt envisagé des moteurs thermiques en 2035 -pour réduire nos émissions de CO2 vont, de leur côté, accélérer cette transition.

vaudrait débattre de sa souveraineté économique et de sa capacité à projeter une économie décarbonée. Voilà nos deux grands enjeux.

coup » -, même si elles peuvent être intéressantes dans le cadre de France Relance, ne suffisent pas. Nous avons besoin de stratégies de filière, de plans de filière négociés entre industriels, syndicalistes et puissances publiques, nationales et régionales,

par une désindustrialisation, par la destruction de l'appareil productif et par un chômage de masse. Chaque fermeture d'entreprise est une épreuve très dure pour les salariés, pour leur famille et pour tous ceux qui, depuis des années, travaillent sur ces sites industriels. Depuis 2017, l'engagement du Gouvernement en faveur de la réindustrialisation est constant. L'État se tiendra toujours aux côtés des salariés pour faire en sorte qu'ils puissent garder leur emploi, pour faire valoir leurs compétences, qui sont exceptionnelles, et pour développer la formation. Le développement du bassin d'emploi doit offrir des perspectives à chacun : aux salariés et à leur famille. Par ailleurs, nous ferons tout notre possible pour débloquer les fonds

Le Gouvernement a donc décidé de faire de la santé l'industrie la plus souveraine et la plus innovante en Europe. Tout d'abord, nous avons tout mis en oeuvre pour soutenir les projets industriels participant à la lutte contre la covid-19. Dès le printemps 2020, nous avons identifié et soutenu les entreprises susceptibles de produire les traitements et vaccins en France. C'est grâce à cette anticipation et à la mobilisation des industriels que plus de 150 millions de doses sont sorties des lignes de production françaises en 2021. En juin 2020, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour renforcer nos capacités de production de médicaments, de traitements, de vaccins ou de composants utiles dans la prise en charge des patients atteints de la Enfin, en septembre 2020, nous avons lancé le plan France Relance, au sein duquel la santé occupe une place centrale. L'objectif est de soutenir l'investissement et la modernisation des industries de santé et de relocaliser les productions. Le plan Innovation Santé 2030, annoncé par le Président de la République en juin dernier, et repris dans le plan France 2030, tire les leçons de la crise sanitaire et fixe la nouvelle ambition de la France : devenir la première nation européenne en matière d'innovation et de souveraineté dans la santé.

vue d'améliorer l'attractivité de la France et la compétitivité de nos entreprises : baisse des impôts de production, réduction de l'impôt sur les sociétés, stabilisation du crédit d'impôt recherche ... La parole

Pour mémoire, en octobre 2018, à la veille du déclenchement du mouvement des gilets jaunes, ces prix avaient atteint respectivement 1,55 et 1,58 euro. Cette hausse entraîne des conséquences particulièrement fortes dans les territoires ruraux,

Ainsi, en Lozère, il faut souvent faire une ou deux heures de route pour se rendre à l'hôpital ou même à la maternité la plus proche. En 2018, alors qu'émergeait le mouvement des gilets jaunes, mon groupe avait déjà proposé un dispositif de minoration de la taxe sur les produits énergétiques dans les départements les plus ruraux.

pour renforcer le pouvoir d'achat des Français. Je pense à la revalorisation de la prime d'activité de 100 euros au niveau du SMIC, à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qui peut être versée jusqu'au début de l'année 2022, à la réduction de l'impôt sur le revenu des classes moyennes ou encore à la suppression de la taxe d'habitation.

Le pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages a progressé de façon continue depuis 2017 et, comme je l'indiquais voilà quelques instants, de 8 % en moyenne sur le quinquennat. Quel que soit leur niveau de revenu, les Français ont bénéficié des mesures fiscales et sociales de ce quinquennat. Un salarié au SMIC peut ainsi gagner 170 euros de plus par mois.

réseau France Services, que conduit Jacqueline Gourault, le Gouvernement fait en sorte que chaque Français ait accès à un point de contact physique et humain à moins de trente minutes de chez lui.

l'attractivité de notre pays est pourtant indéniable si l'on prend comme indicateur les investissements étrangers en France, notamment en raison de la qualité de notre main-d'oeuvre et de sa productivité. En En revanche, ni l'approche financière ni l'idée d'un retour rapide sur investissement ne fondent une stratégie économique de moyen et de long terme. Je rejoins mon collègue Franck Montaugé, lorsqu'il évoque la nécessité d'une montée en gamme de nos produits et services, dans une démarche de développement durable et décarboné, pour Il faut aussi affirmer une volonté d'autonomie, voire d'indépendance stratégique, française et européenne forte, en particulier dans le domaine du numérique, qui transforme nos économies. Le retrait de Scaleway du projet Gaïa-X traduit l'échec l'échec d'un vraiment européen. En France, l'idée d'un souverain a été abandonnée et nous voilà désormais réduits à un de confiance, qui repose sur une base technologique largement Gafam. Il ne suffit pas de financer des start-up, encore faut-il permettre aux infrastructures numériques et aux acteurs concernés de se développer. Monsieur le ministre, le Gouvernement entend-il s'engager réellement dans une stratégie de souveraineté numérique avec les acteurs européens et réduire,

? La parole est à M. le ministre délégué. Madame la sénatrice Blatrix Contat, l'autonomie stratégique dans le domaine du numérique est un enjeu majeur du XXI siècle. L'autonomie de la France et de l'Union européenne dans un monde de plus en plus digitalisé dépendra de plusieurs capacités clés. Premièrement, de notre capacité à maîtriser les technologies critiques du numérique d'aujourd'hui, comme le et l'intelligence artificielle, ou de demain, comme le calcul quantique. nous avons lancé de nombreuses stratégies d'innovation : quantique pour 1,8 milliard d'euros, intelligence artificielle pour 2 milliards d'euros, pour 2 milliards d'euros et cybersécurité pour 800 millions d'euros. En outre, le plan France 2030 viendra renforcer nos capacités de développement dans les secteurs stratégiques.

Troisièmement, de notre capacité à assurer une concurrence loyale et équitable entre les acteurs européens et non européens, entre grandes plateformes et petits acteurs innovants. C'est tout le sens de l'action de la France, qui milite sans relâche pour un marché du numérique régulé et harmonisé à l'échelon européen.

la puissance économique d'un pays se mesure aussi à sa capacité à sécuriser ses débouchés à l'extérieur, notamment dans des secteurs aussi sensibles que la défense ou l'armement. Cela est encore plus vrai dans un monde complexe et multipolaire où de nouvelles puissances émergent et où les relations de confiance s'effritent. Nous en avons malheureusement fait les frais, en septembre dernier, quand l'Australie a unilatéralement décidé de rompre le contrat qui la liait à la France pour la fourniture de sous-marins nucléaires à hauteur de 55 milliards d'euros. Les exemples sont légion et nous incitent à renforcer notre intelligence économique au-delà de nos frontières. Les États-Unis, la Chine, la Russie et tant d'autres sont à l'offensive pour conquérir des marchés hors de leurs frontières et structurer les filières industrielles sur leur territoire. Nous devons faire preuve de réalisme et user de notre influence pour enlever ces marchés, car ces luttes d'influence menacent la puissance économique de la France

Là où d'autres pays, comme l'Allemagne, par exemple, chassent en meute, la France ne joue pas assez collectif. Monsieur le ministre, comment le Gouvernement compte-t-il faire gagner l'équipe de France à l'extérieur ?

Premièrement, il faut renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie. Nous nous y employons en baissant l'impôt sur les sociétés et les impôts de production, en réduisant les charges sur les bas salaires, en menant des chantiers de simplification administrative, en formant de nouvelles compétences ou encore en réformant le droit du travail. ces efforts paient : la France est devenue le pays européen le plus attractif en matière d'investissements étrangers. Deuxièmement, le principe de réciprocité doit s'appliquer à nos partenaires commerciaux. Il est inacceptable que des géants du numérique paient beaucoup moins d'impôts que nos ETI et PME, qu'une entreprise étrangère puisse bénéficier de subventions massives dans son pays pour ensuite gagner des parts de marché en Europe, qu'un État étranger puisse fermer ses marchés publics à nos entreprises, tout en ayant accès aux nôtres. accès aux nôtres. Le Gouvernement se bat pour obtenir une réforme de la fiscalité internationale et soutient les initiatives européennes comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou le projet de règlement sur les subventions étrangères ou en faveur de la réciprocité dans les accès aux marchés publics. Enfin, en ce qui concerne la protection du patrimoine industriel français, critique pour la sécurité nationale, le Gouvernement a renforcé à plusieurs reprises le contrôle des investissements étrangers en France. D'abord, en élargissant, dans la loi Pacte, les secteurs qui y sont soumis ; ensuite, en abaissant de 25 % à 10 %, de

par des normes françaises et européennes. Les pouvoirs publics doivent recourir au prestataire le plus performant et le moins coûteux, indépendamment de sa nationalité. En revanche, si les conditions de concurrence et de réciprocité ne sont pas garanties, alors nous devons intervenir. C'est par la réciprocité que nous parviendrons à soutenir nos industries et à redresser notre balance commerciale, pas par le protectionnisme. En conclusion, la puissance économique de la France passe par un commerce extérieur fort, lequel doit reposer sur l'attractivité du territoire et sur la réciprocité dans les échanges.

consécutives à la pandémie, mettent en exergue certaines failles persistantes de notre économie, qui ont des conséquences sur le financement de la protection sociale et sur l'amélioration du pouvoir d'achat.

d'environ 210 milliards d'euros sur douze mois. En 2021, les exportations françaises devraient avoisiner 470 milliards d'euros contre près de 1 300 milliards d'euros pour les exportations allemandes, soit un écart de 177 % alors que la différence de PIB entre nos deux pays n'est que de 34 %. Certes, nos économies sont différentes, mais cette situation nous enseigne qu'il faut agir sur trois leviers. Tout d'abord, pour vendre plus, il faut produire davantage. Notre voisin d'outre-Rhin peut ainsi s'appuyer sur un formidable tissu de PME, à la fois dynamique, résilient et technologique. Si des mesures ont été prises pour rendre nos entreprises plus compétitives, il faut aller encore plus loin. Ensuite, pour vendre plus, il faut conquérir les marchés là où ils se trouvent, en étant au plus près de la demande. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur notre formidable réseau diplomatique et sur la diaspora, dont j'ai pu mesurer les atouts et le dynamisme lorsque j'étais en charge des Français de l'étranger au ministère des affaires étrangères. Mais cela implique aussi d'augmenter les moyens alloués

La question de l'amélioration de la balance commerciale va de pair avec celles de la réindustrialisation des territoires, de la compétitivité des entreprises exportatrices, de l'orientation géographique de nos échanges ou encore de la montée en gamme de nos exportations. Sur ces problématiques, permettez-moi de rappeler l'action déterminée du Gouvernement, en particulier au travers du volet compétitivité du plan France Relance, d'un montant de 34 milliards d'euros, ou encore du plan d'investissement France 2030, qui ont pour objectif de faire émerger les champions français à l'international dans les secteurs d'avenir. Par ailleurs, nous mobilisons déjà les Français de l'étranger en faveur de notre économie. C'est notamment le rôle des conseillers du commerce extérieur de la France, dirigeants et hauts cadres d'entreprises qui appuient les actions de développement international des entreprises, notamment les PME. Les Français de l'étranger sont également très actifs à travers leurs réseaux locaux, en particulier les chambres de commerce et d'industrie locales, qui jouent un rôle de relais dans 96 pays du monde avec plus de 30 000 membres. à EFE International, structure lancée au printemps 2021, qui permet de recenser les entrepreneurs français de l'étranger et de les associer à la politique de soutien à l'export.

de manière plus qualitative, la crise a conduit nos services économiques et nos ambassades à se rapprocher davantage des Français de l'étranger et de leurs réseaux avec nombre d'actions en partenariat et en solidarité. Ce raffermissement des liens a permis non seulement de soutenir nos compatriotes, qui ont des relations commerciales fortes avec la France, mais aussi de mieux les associer à nos actions locales à destination des exportateurs et des investisseurs. Nous en avons terminé avec